La séance est ouverte. Le compte rendu analytique de la précédente séance a été distribué. Nous n'avons pas reçu. D'observation. Et ce qu'il en a en séance. Je vois point. Le procès verbal est donc adopté sous les réserves d'usage. Madame, la Première ministre, mesdames et messieurs les ministres, mes chers collègues. Notre ordre du jour appelle les questions d'actualité au gouvernement. Notre séance et retransmise en Direct sur Public Sénat et sur notre site internet, chacun sera attentif. Au respect des uns et des autres et au respect du temps de parole. Je ne nie immédiatement la parole au président Claude Malhuret. Pour le groupe les indépendants République. Et Territoires. Chaque jour en Ukraine des femmes et des enfants meurent dans les décombres de leurs immeubles pulvérisés. Chaque jour des soldats tombent. Parce que manque les armes pour résister à Wagner est assez vague d'assaut de traîne misère envoyés au massacre. À Ramstein. Il y a quelques jours, les Européens échoué à s'accorder sur la livraison de chars lourds. Immense déception qui a cédé la place aujourd'hui même à un immense soulagement. L'accord des Allemands, pressé par l'Europe de l'Est et du Nord pour livrer les Léopard de. La France est désormais devant ses responsabilités. Après l'Angleterre, la Pologne, les pays baltes et maintenant l'Allemagne va-t-elle fournir les armements capables de changer l'issue de la guerre. Les chars et une défense sol-air efficaces. Le président de la République, expliqué que ces armements ne doivent pas être escalatoire. La décision allemande dissipe cet argument peu pertinent. On ne peut dire aux Ukrainiens qu'on les soutiendra jusqu'à la victoire finale et en même temps qu'on ne veut pas d'escalade. Parce que par définition la victoire nécessite une escalade depuis un an, nous laissons à Poutine le monopole de l'escalade. C'est lui qui fixe les lignes rouges et nous qui craignons de les franchir alors qu'à chaque franchissement ces menaces sont suivies d'aucun effet. Parce que la Russie est déjà au maximum de ses possibilités. Quant au chantage à l'arme atomique, il est balayé. Depuis qu'à Samarcande qui est maudit ont interdit à un Poutine pétrifiée de s'en servir. Il ne peut plus être l'excuse de nos indécision. Au bout d'un an de guerre. Nous savons que si le coût du soutien à l'Ukraine est élevé. Le coup de ne pas chasser la Russie le serait bien plus. Le but de Poutine n'est pas la seule. Destruction de l'Ukraine. Mais la fin de l'ordre européen démocratique. Il ne s'agit plus d'aider l'Ukraine à se défendre mais a gagné. Madame, la Première ministre. Au-delà des efforts déjà accomplis. Le gouvernement français compte-t-il se joindre à nos alliés et livré l'armement lourd indispensable et quand compte-t-il le faire chaque jour de retard est un jour de deuil en Ukraine. Pour vous répondre. La parole est à madame la Première ministre. Cela fait désormais 11 mois que la Russie a lancé une offensive injustifiable. Inacceptable et brutal sur le territoire ukrainien. 11 mois de bombardements de morts et de drames insupportable pour le peuple ukrainien. 11 mois que l'Ukraine résiste de manière héroïque. 11 mois que la France lui apporte un soutien sans faille. Et comme l'a répété le président de la République il y a quelques jours, nous serons au rendez-vous pour aider l'Ukraine jusqu'à la victoire. Depuis bientôt un an. L'Ukraine peut compter sur l'aide militaire internationale. Aux côtés de nos partenaires, la France s'en prend une part importante. Nous en sommes un des premiers contributeurs par la livraison d'équipements de munitions et la formation de centaines de soldats ukrainiens. Les matériels que nous livrons font la différence sur le terrain, les Ukrainiens le Sunil soulignent eux mêmes régulièrement, je pense aux canons Caesar au système de lance-roquettes unitaires au système de défense aérienne anti- aérienne Crotale livré en fin d'année. Nous entendons les demandes du président et du gouvernement ukrainien. Rien n'est exclu et nous sommes mobilisés pour les soutenir dans la durée. Nous voulons une action coordonnée avec nos partenaires internationaux et qui répondent au mieux aux besoins de l'Ukraine pour assurer sa défense. Pour notre aide militaire. Nous voulons respecter 3 principes. Le premier, comme l'a indiqué le président de la République, c'est que notre aide ne doit pas provoquer d'escalade. Personne n'y aurait à gagner et surtout pas l'Ukraine. Le second c'est que notre aide doit être utile et efficace rapidement. Cela implique notamment que les forces ukrainiennes soit en mesure d'être formés pour utiliser les équipements et qu'elle puisse en assurer le maintien en condition opérationnelle. Enfin, nous ne devons pas et nous ne pouvons nous ne voulons pas affaiblir significativement nos propres capacités de défense en particulier les plus critiques. Je salue la décision de l'Allemagne sur le sujet des chars lourds, elle permettra de renforcer les capacités militaires ukrainiennes en matière de combat blindés. Nous avons été particulièrement réactifs aux demandes de l'Ukraine en la matière. Début janvier, le président de la République avait initié une dynamique en annonçant la livraison de chars légers AMX 10 RC. La décision allemande renforce et amplifie le soutien engagé. S'agissant des chars Leclerc nous poursuivons l'analyse avec le ministre-désarmer la question de l'aide à l'Ukraine ne se limite pas à tel ou tel équipement. Chaque pays dispose de domaines d'excellence comme la défense aérienne et l'artillerie pour la France et il est important de bien nous coordonner. Enfin j'ajoute que nous avons créé un fonds spécial de soutien de 200 millions d'euros pour permettre à l'Ukraine d'acheter le matériel dont elle a le plus besoin directement auprès de nos industriels. Nous sommes également actifs au niveau européen en prenant toute notre part à la Facilité européenne pour la paix. Monsieur le Président Maluret, vous le savez, j'avais eu l'occasion de le rappeler lors du débat qui s'était tenue le 26 octobre. Ici même notre soutien à l'Ukraine dépasse le seul cadre militaire, c'est aussi un soutien humanitaire diplomatique. Un soutien grâce aux sanctions sans précédent de l'Union européenne contre la Russie et un soutien bien sûr à la reconstruction du pays. Nous agissons en lien constant avec nos partenaires européens et nos alliés. Nous agissons avec détermination et constance. Nous serons aux côtés de l'Ukraine jusqu'au bout. Je peux vous l'assurer. Je vous remercie. Merci madame, la Première ministre. La parole est maintenant notre collègue Philippe Tabarot pour le groupe Les Républicains. Merci monsieur le président, ma question s'adresse à Madame, la Première ministre madame, la Première ministre. Les classes moyennes ne croit plus et n'écoute plus, ce qui les dépossède. C'est en ces termes, Si jusque le géographe Christophe Guilluy s'exprimer cette semaine dans un grand quotidien. C'est une illustration parfaite du ressenti des Français à la mise en place forcée des zones à faibles émissions mobilité notre groupe ici au Sénat, l'a rappelé il y a quelques jours lors d'un débat que nous avons souhaité, après la mise en place chaotique des ZFE du Grand Paris à Toulouse en passant par Strasbourg, Nice ou Toulon. Nous y avons défendu une vision équilibrée entre le tout voiture que nous récusons, et le jusqu'au-boutisme environnementales qui voudrait supprimer tous les véhicules. Les Français sont-ils informés que 40% d'entre eux vont devoir, dans les prochaines années amener leur véhicule à la casse. Non. L'industrie automobile française, et je dis bien française est-elle prête à cette transformation vers le tout électrique. Non, d'après Monsieur Tavarès l'avitaillement est-il suffisant et l'impact de la crise énergétique intégrée au cou et au déploiement des bornes électriques non. La logistique urbaine est-elle organisée pour nos petits artisans et leurs véhicules utilitaires. Non. Les contrôles sont-ils efficaces et efficients. Non. L'offre de transport en commun enfin est-elle suffisante ponctuel et Éric-t-elle l'ensemble de notre pays. Non. Les ZFE tels que vous les avez mis en place sont un capharnaüm, tout est à l'envers madame, la Première ministre, avez-vous conscience que ces ZFE pourrait être l'étincelle de nouveaux blocages allez vous mettre fin à cette marche forcée en sens inverse. Pour vous répondre. La parole est au. De la. Transition écologique et de la cohésion des territoires monsieur Béchu. Monsieur le président. Mesdames, et messieurs les sénateurs, Monsieur le Sénateur Tabarot. Y a-t-il ici des gens qui pensent que la question des décès par la pollution atmosphérique est un sujet secondaire. Y a-t-il ici des gens qui contestent la nécessité de lutter contre le dérèglement climatique. Y a-t-il ici des gens qui considèrent qu'il faut faire confiance aux élus locaux. Quand on met en place des politiques. Eh bien Mesdames et messieurs les sénateurs, Monsieur le Sénateur Tabarot. Vous avez dressé la feuille de route qui est la nôtre. Les zones à faibles émissions. Salut. Les zones à faibles émissions de quoi s'agit-il. D'une invention française non. Ça existe dans 14 pays d'Europe. La première a été mis en place en 1996 en Suède. Est ce que ce dispositif concerne 40% des automobilistes non. Il concerne. Les agglomérations qui sont en dépassement de seuil à la suite de la condamnation par la Cour de justice des Communautés européennes et par le Conseil d'État le seul calendrier fixé par l'État. Je n'ai aucun doute sur le fait que vous voulez rassurer nos concitoyens et faire en sorte que nous prenions les bonnes décisions. Je vous demande juste d'entendre ce qu'est l'état du droit, l'état du droit, c'est qu'il n'y a pas de calendrier. Fixé par l'État par rapport aux véhicules professionnels. L'état du droit, c'est que les seuils de restrictions dépendent des dépassements de la pollution de l'air et qu'à la minute où nous nous parlons, contrairement à ce que certains disent c'est ni tout le pays ni 43 agglomérations qui sont concernés par un calendrier restrictif le seul calendrier restrictif fixé par la loi, c'est la sortie des critères cinq si vous êtes en dépassement de seuil au 1er janvier 2023. Critères IV au 1er janvier 2024 critères, 3 au 1er janvier 2025. Combien avons-nous aujourd'hui d'agglomération dépassement de seuil. On en a moins de 10. Les autres, elles ont à la fois une attitude sur la mise en place de mesures qui permettent d'atteindre les objectifs puisque c'est une obligation. De résultat pas une obligation de moyens. Les critiques que vous avez mise et dont je me suis réjoui dans cet hémicycle et qui était à la fois plus nuancé plus constructive que le caractère commencer de la question. Elles nous ont conduit à mettre en place un groupe de travail qui associe qui. La métropole de Toulouse et celle de Strasbourg au cours proposer des solutions. Faut que c'est l'état d'esprit du gouvernement. gouvernement. Madame, la Première ministre. Je regrette votre absence de réponse car c'est vous qui avait également souhaité comme ministre des Transports à l'époque, ces ZFE. Écoutez, s'il vous plaît, accompagnez nos concitoyens pour que les ZFE ne devienne pas un sacrifice de plus pour les Français. La parole est à notre collègue Stéphane Demilly pour le groupe de l'Union centriste de la parole. Merci monsieur le président. Ma question s'adresse directement à Monsieur le Ministre du Travail et indirectement à tous ceux qui aiment la démocratie. Les semaines passent et avec elles s'approche un projet de loi que personne ne peut ignorer tant il est médiatisé tentent il déchaîne les passions et tant il est vrai il impactera la vie future de nos concitoyens. Je parle naturellement de la réforme des retraites. Certains le soutiendront sans réserve d'autres l'amenderont pour le rendre plus conforme à leurs convictions. D'autres enfin le combattront fermement. Les avis divergeaient parfois au sein d'un même groupe parlementaire. Mais là n'est pas l'objet de mon intervention, car nous aurons naturellement l'occasion de revenir sur ce sujet en février lors des débats. Je souhaite plutôt vous parler de la forme et du climat qui prévaut à ses futurs échanges. La semaine dernière. Un important responsable syndical a déclaré, je cite qu'il allait s'occuper des élus qui soutiendrait ce texte en organisant des coupures de courant les ciblant directement. Je trouve ces propos terriblement scandaleux. Dans une démocratie, on peut et on doit débattre les orientations politiques. On peut les soutenir. On peut les critiquer, on peut naturellement manifesté en revanche menacé un élu, parfois même dans sa vie privée pour ses prises de position ce n'est pas tolérable. En démocratie, c'est la force des arguments qui compte et non les arguments de force. La réflexion, l'écoute, la sérénité et au final, le jugement ne doivent pas être à la merci de toute forme d'intimidation, de pressions ou de menaces. Tous les bancs de cet hémicycle devrait dénoncer de telles méthodes barbares. Monsieur le Ministre, comment comptez-vous ramener de la sérénité et de la lucidité dans ce débat budgétaire et sociétal dont tout le monde gagnerait à ce qu'il soit beaucoup plus apaisée et beaucoup plus constructif. On vous répond de la parole est au ministre du Travail, du plein emploi et de l'insertion, monsieur Dussopt. Merci monsieur le président, Mesdames, et messieurs les sénateurs, Monsieur le Sénateur demi-. À vrai dire, je partage tout et je crois que nous sommes nombreux ici sur les bancs du gouvernement et j'imagine aussi sur les bancs du Sénat à partager votre intervention et à partager votre indignation. Le débat sur les retraites est ouvert et c'est effectivement un débat qui peut être vif, un débat qui peut être invité. Un débat qui peut être passionné et je n'ai aucun doute sur le fait qu'à l'Assemblée nationale comme ici, nous aurons ces débats-là. Avec la Première ministre. Nous souhaitons que ces débats soient les plus constructif possible. Le plus ouvert possible et nous sommes convaincus que. Cette capacité à mener le débat de bonne qualité jusqu'au bout, passe à la fois par l'affirmation de conviction et l'affirmation de priorité. Les notes sont l'équilibre du système sont la protection des plus fragiles sont les mesures les plus justes pour accompagner la mise en oeuvre de réformes qui doivent justement nous permettent de revenir à l'équilibre du système et ainsi de le pérenniser. Dans le cadre de ce débat des mouvements sociaux sont organisées et les organisations syndicales sont légitimes, a appelé à des mouvements de grève ou à des mobilisations elles sont toutes aussi légitimes à le faire lorsque les choses se passent bien comme elles se sont bien passées dans les cortèges de la semaine dernière. Mais dans ce débat-là. Nous l'avons dit aussi nous ne souhaitons ni blocage Qui serait pénalisant pour l'ensemble des Français et nous n'acceptons aucune menace les propos que vous avez évoqué, ce ne sont pas acceptables et un certain nombre des propos qui ont été tenus. Des actions qui ont été envisagées si elles étaient réalisées relèveraient du délit plus que de l'action politique ou de l'action militante et donc nous serons sur cette ligne-là, à la fois de clarté d'affirmation de conviction mais avec le souci permanent de veiller à ce qu'aucun acte inacceptable ne puisse être commis au delà de votre question, monsieur le sénateur, et au-delà de ce contexte autour de la réforme des retraites. Ces menaces proférées à l'encontre d'élue pour les convictions qu'ils expriment les positions qu'ils prennent ne sont vie évidemment pas acceptable et renvoie un autre contexte qui est celui de l'augmentation des faits de violences contre les élus. Et votre question me permet, je le dis sous le contrôle du ministre de l'Intérieur de souligner qu'aujourd'hui même au Journal officiel a été publié la loi qui autorise les associations d'élus et les assemblées parlementaires à se porter partie civile aux côtés des élus qui ont été victimes de violences. C'est aussi un progrès qu'il faut souligner pour bien protéger les élus français. Je donne la parole à notre collègue Cathy pour se polie pour le groupe communiste, républicain, citoyen et écologiste avait la parole. Merci monsieur le président. Monsieur le ministre du Travail. Évidemment si vous reportez l'âge légal à 64 ans, elles sont un peu plus pénalisés sur ce point là elles sont un peu plus un paqueté que les hommes et syndicalistes, un opposant à votre réforme des retraites qui a tenu ces propos. Non. Cette réalité, des conséquences de votre réforme des retraites, c'est le ministre Riester qui le reconnaît. Vous ne pouvez pas dire que ce sont des mensonges avec votre réforme, les femmes vont devoir en moyenne travaillé 7 mois de plus pour partir en retraite, contre 5 mois supplémentaires pour les hommes. Cette réforme profondément injuste pour l'ensemble des salariés. Il est encore plus pour les femmes. Votre réforme va donc aggraver les inégalités entre les femmes et les hommes. Commencer plutôt par imposer l'égalité salariale entre les femmes et les hommes pour dégager 6 milliards de cotisations de retraite supplémentaire. Je pense à ces ouvrières à ses ouvriers de la marée de Boulogne au travail dès 2h du matin à celles et ceux des industries agro-alimentaires debout derrière leurs chaînes toute la journée, qui ont commencé leur carrière tôt ces travailleurs vont cumuler tous les aspects négatifs de votre réforme. Je pense aux aides à domicile aux soignantes aux infirmières aux femmes de ménage aux caissières que vous applaudit. Durant la crise sanitaire qui devront travailler neuf mois supplémentaires pour les générations de 1972 à l'issue du conseil de ministres. Vous avez reconnu Monsieur le Ministre, que le recul de l'âge légal. Serait plus favorable aux femmes qu'aux hommes dans un 1er temps. Par vos propres aveux, vous établissez l'injustice de votre texte. Nous vous demandons de le retirer et d'organiser un véritable débat dans le pays. Pour vous répondre. La parole est au ministère du Travail, du plein emploi et de l'insertion, monsieur Dussopt. Si. Merci monsieur le président, madame la sénatrice. Alors si Paulo. Quelques mots pour revenir sur les faits que vous évoquiez sur la lecture, qui peut être fait parfois ici ou ailleurs d'ailleurs de l'étude d'impact qui accompagne le projet de loi de réforme des retraites. Peut être en rappelant quelques. Évidences mais qu'il vous faut rappeler dans un tel débat. Est-ce que l'âge d'ouverture des droits sera différent entre les hommes et les femmes, non. Est-ce que la durée de cotisation requise entre les hommes et les femmes portera une différence évidemment non. quelles sont les conséquences de la réforme que nous portons. Il y a effectivement un rapprochement de l'âge effectif, je ne parle pas de l'âge légal mais de l'âge effectif de départ entre les hommes et les femmes. Mais vous l'avez certainement noté Madame la sénatrice à la lecture de ce rapport d'évaluation en 2030 les femmes continuera à partir plus jeune que les hommes à la retraite et pourquoi elles pourront continuer à partir plus jeune que les hommes à la retraite parce que nous maintenons l'intégralité de ce que nous appelons les droits familiaux. Les quatre trimestres automatiquement attribuée aux femmes, à l'occasion d'une maternité c'est quatre pour le régime général de pour le régime de la fonction publique et vous savez que dans le régime général, il y en a 4 qui peuvent être répartis librement entre les membres du couple. Vous avez aussi vu madame la sénatrice dans ce même rapport d'évaluation que les mesures que nous prenons en matière d'éligibilité à la retraite minimale garantie comme en matière d'éligibilité au départ anticipé au bénéfice des carrières longues sont favorables aux femmes parce que nous intégrons les codes et trimestres cotisés au type de l'assurance vieillesse des parents au foyer dans les trimestres requis pour déterminer cette éligibilité tant au minimum de pension qu'au dispositif de départ anticipé pour carrière longue. Nous avons veillé scrupuleusement avec un chef du gouvernement dans chacune des décisions que nous avions apprendre à protéger les plus fragiles. Tous les exemples que vous avez cité tous les métiers que vous avez évoquées, font partie de ceux qui seront mieux protégés et mieux accompagner tant par les dispositifs de pénibilité que par le nouveau dispositif de prise en compte des carrières longues pour ceux qui ont commencé à travailler avant 18 ans, je suis sûr que dans le débat, nous trouverons des convergences sur ces points là. On a ma force polie pour quelques secondes. Monsieur le Ministre, vous avez refusé l'étude d'impact. Vous êtes incapables aujourd'hui de nous donner le nombre de Françaises qui est de français d'ailleurs Monsieur le mini et s'il y a 10 ans, vous êtes chez le grand défenseur de la retraite à 60 ans vous avez changé évidemment Davy entre deux, mais ce n'est pas étonnant de votre part. La parole est notre collègue Ludovic et pour le compte du Rassemblement des démocrates, progressistes et indépendants. Monsieur le président, Mesdames, et messieurs les ministres, mes chers collègues, ma question s'adresse à monsieur Sébastien Lecornu Ministre des Armées. Monsieur le Ministre, le 20 janvier dernier lors de la présentation de ses voeux aux armées à Mont-de-Marsan. Le président de la République a indiqué que la France a louerait à ses armées un budget davantage conséquent sur la période 2024 2030. La prochaine loi de programmation militaire articulée autour de 4. Pivot principaux, à savoir notre coeur de souveraineté la haute intensité. La protection de nos intérêts et nos partenariats renouvelé. Attribuera 413 milliards d'euros aux forces armées, soit 118 milliards de plus que la loi de programmation militaire actuel même s'il convient de tenir compte d'un présent contexte inflationniste. Le président de la République a rappelé le contexte particulier de menaces dans lequel nous sommes et l'émergence des formes de conflictualité nouvelle. Cet effort conséquent rassure non seulement notre communauté militaire nos décideurs et nos élus. Mais également notre communauté et qu'il traduit de faire de la, du président de la France, un président plus souverain plus entreprenants et plus Agile. Cet effort ne permettra indubitablement d'avoir une guerre d'avance notre Parlement y veillera. Notre souveraineté passera non seulement par le renfort de notre dissuasion par nos postures permanentes mais aussi par la résilience nationale. Il est vrai qu'il nous faut agir partout plus vite et plus fort. Cette dernière LPM placée sous le signe de la transformation prendra le relais de l'ancienne qui avait déjà été marqué par un effort significatif en matière de réparation. Cela demandera assurément une forme et d'agilité car comme vous le savez. De nombreuses infrastructures dépendent totalement du matériel qu'elle supporte. Je pense notamment aux bases aériennes exclusivement équipés de d'avion de type Mirage. Ou d'établissements de type CIA qui maintiennent aujourd'hui des hélicoptères d'ancienne génération de type Gazelle ou type Puma et qui peine à se projeter dans l'avenir. Monsieur le Ministre, dans un contexte où la souveraineté est redevenu un axe de réflexion important de tout 1er plan, comment pensez-vous concilier cette politique forte de transformation. Avec le développement de nos infrastructures militaires et de notre industrie de défense de nos territoires. Monsieur le ministre, conclure. Comment souhaitez-vous associer les territoires à cet effort inédit sans égal mesure depuis la présidence du général De Gaulle. Pour vous répondre. La parole est au ministre des armées, monsieur Sébastien Lecornu derrière. Si Monsieur le président du Sénat, Mesdames, messieurs les sénateurs, Le ministère des Armées est un grand ministère territorial et pour cause, il est représenté présents dans les différents territoires et donc de fait. En deux minutes, lister les impacts de la programmation militaire est très difficile. Je vais essayer de donner quelques lignes bon hein déjà la réparation continue c'est particulièrement vrai sur les infrastructures, on le sait très bien beaucoup de régiments beaucoup de base navale beaucoup de bases aériennes sont encore dans un état absolument déplorable, fruit de décision qui parfois ont été prises il y a très longtemps et sur lequel la réparation il faut donc le dire avec humilité. La 2ème des choses la réparation continue sur les services de soutien. C'est particulièrement vrai pour le commissariat. C'est vrai pour le service de santé des armées. Je sais que c'est un sujet qui est suivi par les membres de la commission de la Défense et des forces armées du Sénat et là on le voit bien ses soutiens aussi ont été abîmé la réparation prendra du temps dans des contextes qui sont difficiles, alors c'est quand on parle de transformation. Il va sans dire que ces transformations vont être moins spectaculaire sur les territoires que dans le passé et pour cause, déjà parce qu'on ne ferme aucun régiment aucune base aérienne où aucun laboratoire de la DGA, donc par définition c'est une transformation interne. Ah Babouri. C'est vrai sur le terrain technologique. Vous l'avez cité le scorpion rafales. Il y a des sauts technologiques, qui sont importants et qui vont forcément transformer la vie des unités. C'est vrai également sur les métiers nouveaux, le cyber le spatial. Les fonds sous-marins. On aura l'occasion d'y revenir, ici même, c'est vrai également aussi pas Transformation RH du du ministère puisque vous aurez forcément un pivot en matière de ressources humaines liées soit aux réserves avec un nouveau ratio de réserves, il sera un impact important pour les régiments de l'armée de terre et dans le Grand-Est, singulièrement, on sera amené à y revenir dans les temps qui, qui viendront. C'est vrai aussi pour le pyramidal entre les sous-officiers et la troupe puisque les fonctions nouvelles qui amène ce saut de technologie demande aussi évidemment beaucoup plus de de savoir-faire en tout cas une montée en puissance de compétences, je reviendrai vers vous sur ces sujets, on peut aussi citer en 10 secondes l'impact en matière d'emploi pour la abbaye. Aux 4 coins de l'Hexagone une feuille de route pour l'outre-mer que le président de la République vaudra détaillé lui-même sur les impacts de loi de programmation militaire pour nos territoires ultramarins et la relation avec les collectivités territoriales sur lequel je veux qu'on arrive à systématiser les choses, notamment pour le plan famille. Merci monsieur le sénateur. Je vais donner la parole maintenant à la. Présidente Laurence Rossignol. Pour le groupe socialiste. Écologiste et. Merci monsieur le président. Lundi le Haut Conseil à l'égalité a rendu son rapport. Ce rapport confirme la persistance du sexisme à haut niveau dans notre société, ce qui explique d'ailleurs que la condition des femmes reste soumise aux inégalités et aux violences cet écosystème sexistes impose aux femmes de tous toujours devoir s'adapter. Et ce qui v résister. C'est un effort constant et puisqu'on parle d'effort. Le même jour avec un sens du timing. Étonnant le ministre Riester dans un moment de franchise. Merveilleux, a dit en effet, cette réforme va demander aux femmes un effort supplémentaire. Alors je dis clairement pour ce qui est des femmes, les efforts c'est non, on en fait déjà assez comme ça tout le temps. Vous répétez en boucle que la pension minimum va passer maintenant à 1200 euros. Mais les conditions d'accès à cette pension, celle d'une carrière complète sont tellement drastiques que justement elles vont éviter les femmes, les femmes justement ont des carrières hachées, elles ne pourront pas profiter de cette, de cette pension à 1200 euros, dont vous nous parlez. Par ailleurs, il y a une chose qui est sûr c'est qu'elles vont devoir travailler plus longtemps et non seulement plus longtemps mais plus longtemps que les hommes qui vont devoir travailler plus longtemps puisque selon les études des experts. Ce sera le double d'un allongement de la durée du travail pour les femmes à à partir de 1972, c'est un peu compliqué, mais ça prouve quand même que votre réforme accroît les inégalités entre les femmes et des hommes comme toutes les réformes qui sont supposés être neutres et qui en réalité accroissement les inégalités. Alors puisqu'on parle d'effort, les femmes en font beaucoup, je l'ai déjà dit madame, la Première ministre vous vous pouvez en faire hein. Vous êtes la femme qui peut faire un bel effort en renonçant à cette retraite injuste pour les femmes. On vous répondre. La parole est au ministre du Travail. Il plaide emploi de l'insertion. Merci monsieur le président, madame la présidente Rossignol. Je ne reviens pas sur les les éléments que j'ai donné en réponse à Madame. La sénatrice du groupe communiste précédemment. Simplement vous dire un certain nombre de choses. La réforme que nous menons est une réforme qui porte des protections pour les femmes. Vous avez du mal à l'entente je crois ou à le concevoir mais au-delà des dispositions que nous prenons. Il y en a une que je n'ai pas rappelé qui est que nous avons veillé à ce que l'âge de suppression de la décote soit maintenue à 67 ans l'âge de suppression de des Côtes d'aujourd'hui parce que 20% des femmes ont une carrière incomplète et que ce sont l'essentiel des de celles et ceux qui vont jusqu'à 67 ans qui justement sont des femmes. Nous veillons avec la retraite minimum à ce que justement les femmes qui ont les carrières les plus fragiles des carrières hachées que vous avez décrite les carrières avec les revenus les plus bas soit bénéficiaire la retraite minimum que nous mettons en place va permettre à 200.000 nouveaux retraités par an, c'est-à-dire un départ à la retraite sur 4 de bénéficier d'une pension meilleur avec la réforme que sans la réforme et les deux tiers ses bénéficiaires sont des femmes parce que justement et là je vous rejoins, les femmes sont les plus exposés à la précarité et aux carrières agit le le temps me manque pour décrire les mécanismes mais le fait que nous ayons en fait le choix de revaloriser le minimum contributif majoré qui est accessible des 120 trimestres cotisés, le fait que nous ayons fait le choix de revaloriser le minimum le revaloriser le minimum contributif de base accessible à toutes celles et ceux qui ont travaillé permet justement de protéger les plus fragiles. Nous n'avons pas les mêmes priorités Madame la sénatrice. Vous parlez de carrière complète vous parlez de carrière complète. Nous nous adressons justement à celles qui n'ont pas des carrières complètes et qui bénéficieront des revalorisations et des systèmes de protection que nous mettons en place, c'est ça, notre priorité protéger les plus fragiles protéger celles et ceux qui sont exposés à la précarité et aux difficultés, difficultés de carrière c'est avec cette loi que nous allons faire et c'est avec ces dispositions que nous allons-y arriver je termine par un point pour souligner un point d'accord avec votre question, vous avez cité le le rapport du Haut Conseil à l'égalité et ce au Conseil montre aussi que notre système de retraite qu'on accuse parfois tous les mots est aussi le réceptacle d'une vie d'inégalités, travaillons sur ces inégalités, faisant en sorte de les résorber et les retraites seront beaucoup plus juste, tout le monde en sera satisfait. La parole est à notre collègue Henri Cabanel pour le groupe du Rassemblement démocratique et ceci à l'heure. Merci monsieur le président. Monsieur le Ministre de l'Agriculture la souveraineté alimentaire la viticulture et la filière qui a subi le plus d'alerte successifs lundi le président de la Chambre culture de l'Hérault a pris l'initiative d'une réunion en urgence pour alerter les parlementaires de cette crise sans précédent. 2019. Taxe Trump 2022 1021 Covid 2021 énormes, gel de la grêle de la sécheresse. 2022. Guerre en Ukraine avec ses conséquences économiques, au-delà du drame humain, pénurie de bouteilles, augmentation du prix du verre, des engrais, du carton et cetera et l'inflation qui a elle n'aime pas directe sur la consommation par exemple, moins 15% sur les vins rouges. Chiffre très inquiétant car la viticulture française est un secteur qui réalise plus de 14 milliards d'euros d'excédent commercial. Le Bordelais a récemment manifesté sa colère car le désespoir gagne ses vignerons. Nous venons avec le groupe. Avant la séance. Reçu un collectif de viticulteurs bordelais abattu désespérés mais combatifs. Lundi, le président des de l'Hérault, consterné, a souligné la catastrophe du contexte pour les jeunes installés depuis 2 3 ans qui est qui accumule les galères et les crises, alors que leur projet d'Ethical est parfaitement sain. Si une remise en question structurelle est nécessaire et les organismes professionnels par que proposez-vous Monsieur le Ministre pour aider cette filière. Allez-vous se tenir la demande d'étalement de remboursement des PGE de 6 à 10 ans. Allez-vous répondre à la demande de distillation adossé à l'arrachage temporaire ou définitif à l'aide au stockage. Allez-vous soutenir la création d'un plan de relance commerciale. Pour répondre. La parole était. Ministre de l'agriculture de la souveraineté alimentaire monsieur Fesneau. Merci monsieur le président, Mesdames, et messieurs les sénateurs, Monsieur le Sénateur Cabanel, merci de cette question, vous avez raison, la situation dans la filière. Vitivinicole vinicole Elle a commencé ou les premières alertes ont été faites, d'ailleurs votre collègue la sénatrice de la tu m'avait alerté. Dès cet été, elle a commencé en particulier dans le Bordelais. C'est le cumul comme vous l'avez dit de différentes crises, sur lesquelles d'abord je je tiens à le dire, le gouvernement et vous le savez beaucoup intervenue puisque sur le gel, il a couvert à hauteur d'un milliard d'euros la perte qu'il est intervenu aussi sur d'autres dispositifs pour accompagner la filière. Ceci dit, vous avez raison, ça ne suffit pas parce que nous sommes dans une crise à la fois conjoncturelles à une crise structurelle crise conjoncturelle liée à l'augmentation particulier des matières sèches. Et l'liée et poussés par l'inflation des prix du carburant et des produits pardon des matières énergétiques en particulier et donc on on a travaillé sur un plan d'allégement des charges et qui concerne aussi les viticulteurs. Nous devons travailler et nous sommes en train, travaille avec les services tout ce qu'on a sur la table trois ou quatre dispositif le 1er c'est la poursuite du PGE. Nous y travaillons avec le ministère de l'Économie et des finances pour voir dans quelles conditions, ça peut se faire, le 2ème élément c'est l'aide au stockage ou à la distillation. Qui peut être un élément complémentaire pour régler. Le le trop sur les choses et puis le 3ème élément qui est un élément plus structurelle qui est l'arrachage. Je pense en particulier à ce qui se passe dans le Bordelais pour réguler. Une surproduction qui est surproduction structurelle, pour le coup, et puis évidemment, nous devons travailler. Sur ce que vous avez dit, c'est-à-dire la capacité qu'à cette filière a aussi ou s'ouvrir des perspectives à l'export. Il y a une évolution des modes de consommation il faut qu'on puisse en tenir compte et l'ensemble de ces dispositifs qu'on est en train d'expertiser c'est compliqué pour chacun d'entre eux, à la fois pour des raisons budgétaires. Pour le PGE, c'est compliqué aussi pour d'autres raisons dont on a besoin de regarder précisément ce qu'on peut faire et on dira en vérité ce qu'on peut faire et ce qu'on ne peut pas faire aux filières je les réunirai au tout début du mois de février pour regarder l'ensemble des dispositifs et apporter les premières réponses concrètes reconnaissons aussi qu'il y a un certain nombre de dispositifs qui relève du règlement communautaire, je pense en particulier à l'arrachage qui nécessite du temps donc j'ai besoin avec vous et avec eux de construire des mesures d'urgence et puis des mesures qui leur donne des perspectives sur le moyen long terme parce que c'est bien, c'est de tension qu'il faut essayer de de conjurer et aussi en tout cas en particulier pour les jeunes mais pas pas seulement de leur donner des perspectives, parce que la crise est en effet assez grave. Merci monsieur le le ministre de de ses réponses. Vous savez, nous sommes nombreux sur tous ces bancs à vouloir que la France reste la référence mondiale au niveau du vin. Vous l'avez dit, la situation est grave mais et certainement elle est pas désespéré aussi je vous propose donc de vous appuyer sur tous les parlementaires au delà de votre majorité qui connaissent parfaitement leur territoire parce que l'union fait la force et je crois que la viticulture a besoin de ça. Merci. Merci. La parole est à notre collègue Yémen Haroche pour le groupe écologiste solidarité et Thierry. Merci monsieur le président, ma question s'adresse au ministre de la justice et concerne quartier disciplinaire. Ces lieux ne sont pas perçues par hasard comme des lieux de moindre droit les conditions de vie sont plus dur qu'en détention général les garanties comme la superficie minimale des cellules, la possibilité de promenade la possibilité de contact avec l'extérieur par les droits de visite ou par le téléphone semble parfois oublier l'État français de bruit, pas par l'état de ses prisons et par les conditions de détention, les quartiers disciplinaires sur le reflet exacerbé de ces problèmes et le comité pour la protection contre la torture du Conseil de l'Europe. Ah. Lors de sa visite établi de nouveaux des constats qui ne nous font pas honneur actuellement la durée maximale. Il est de 30 jours. Le comité a recommandé à nouveau aux autorités françaises de prendre les mesures législatives nécessaires pour assurer que le placement à l'isolement disciplinaire ne dépasse pas 14 jours pour une infraction donné qu'on puisse parler d'adultes et soit de préférence d'une durée inférieure, ces recommandations nous paraissent nécessaires et le début d'une réelle prise en compte des difficultés au sein des quartiers disciplinaires et je me dois d'évoquer les doutes portés sur les mauvais traitements et le manque de transparence, de traçabilité qui hélas fait croître et les doutes et les suspicions entre autres sur les circonstances de certains événements et de certains suicide suicide qui semble aussi plus important dans ces lieux où les privations peuvent créer des conditions favorables au passage à l'acte, le CPT regrette aussi que le recours à la force qui peut parfois parfois se justifier ne soit pas systématiquement répertoriée et quand il est que les données de permettent pas de démontrer en quoi celui-ci s'avère strictement nécessaire et appliqué dans le le respect du principe de proportionnalité aussi je souhaiterais savoir si le ministère compte rendre disponible les chiffres liés au quartier disciplinaire nombres de séjour durée, durée moyenne d'ombres de suicide afin de permettre à l'état des lieux de la situation et pour enclencher une réforme des quartiers je souhaiterais aussi connaître votre avis sur les possibilités d'aménager les restrictions aux conséquences trop importantes sur les détenus des quartiers disciplinaires. sénateurs, ce sénateur ben Haroche. Je vous communiquerai très volontiers les chiffres, je vais demander à la direction de l'administration pénitentiaire de me les communiquer. Dès que je excuser je voulais communique mais ne laissons pas entendre ou s'il vous plaît que. Le quartier disciplinaire, autrement appelé mitard serait le lieu de l'arbitraire absolu. Je rappelle que. Un détenu quand il est envoyé au mitard comparaît devant une commission composée du directeur de l'établissement pénitentiaire d'un assesseur qui vient de la société civile, qu'il peut être défendu par un avocat. Naturellement, nous avons évoqué ici au Sénat, c'est le président François Noël Buffet qui est à l'initiative de cette. Proposition de loi sur les conditions les conditions indignes, elle touche la détention ordinaires comme naturellement les quartiers disciplinaires et nous y sommes particulièrement sensible je veux à ce titre vous indiquer que nous avons consacré plus de 130 millions d'euros d'euros par an pour la rénovation. Mais les choses ne se font pas en un claquement de doigts. J'ai déjà eu hélas. L'honneur et le déplaisir en même temps de le dire, la justice c'est un abandon. Deux 3 décennies sur le plan humain, sur le plan budgétaire et sur le plan politique. Par ailleurs s'agissant des suicides. Évidemment que le quartier disciplinaire peut être un facteur. Favorisant si j'ose dire. Nous y sommes très attentifs. Le personnel pénitentiaire. Prendre un certain nombre de dispositions. Nous faisons venir des médecins également pour que. On s'occupe davantage des détenus tout cela et tu en cohérence parce que vous avez bien compris que le suicide d'un détenu hein n'échec je vous ouvrent la porte de la Chancellerie je vous communique les chiffres. Monsieur le sénateur très prochainement et nous réfléchirons ensemble à ce que vous avez évoquées, mais je le dis, ça n'est pas pour le moment à l'ordre du jour. Remercie Monsieur le mini je voulais juste signaler que quelques fois certains processus administratifs peuvent créer des problèmes par exemple le passage en quartier disciplinaire de détenus parce qu'ils possèdent des portables qui de 100 pas ce qui sont bien à disposition par l'administration et on sait que les contrats les marchés d'État de l'administration font que ces portables à leurs coûts de communication coûte. 10 fois plus cher que Nep copeaux d'lequel d'entre nous, le coût d'une communication normale. Donc il y a aussi un certain nombre de mesures à prendre, y compris dans des marchés qui sont passés aujourd'hui par l'État et le ministère. Pour ces matériels. La parole est à notre collègue Laure Darcos pour le groupe Les Républicains. Merci monsieur le président, ma question s'adresse à monsieur le ministre du Travail, du plein emploi et de l'insertion. Monsieur le Ministre, le gouvernement vient de présenter sa réforme des retraites et le moins que l'on puisse dire est que les femmes pourraient être les grandes perdantes, des mesures à venir. L'étude d'impact, le démontre clairement. Devront travailler en moyenne sept mois de plus alors que les hommes ne seront astreints qu'à cinq mois supplémentaires. En outre, de nombreuses femmes pouvaient partir dès 62 ans à taux plein grâce au trimestre acquis lors de la naissance de leurs enfants. Avec votre réforme, elles devront travailler 2 ans de plus pour atteint le nouvel âge légal de 64 ans et perdront le bénéfice de cette bonification. Vous aurez beau jeu de souligner qu'en travaillant plus longtemps et bénéficieront d'une retraite revalorisées, vous ne manquerez pas de rappeler également qu'elles seront les premières bénéficiaires de la hausse au minimum de la pension du minimum de pension. Mais de quelle retraite parlons-nous. Vous n'ignorez pas que la retraite des femmes est de 40% inférieure à celle des hommes parce qu'elles sont les premières victimes des inégalités salariales. Vous ne pouvait ignorer non plus qu'elles ont des carrières fréquemment interrompues par des maternités qui réduisent la durée de cotisation et font d'elle les plus touchés par la décote. Dans ces conditions, il est indispensable de compenser l'effort supplémentaire demandé aux femmes de mieux en prendre en compte leur maternité car une réforme des retraites par répartition ne peut se désintéresser de la politique familiale et d'avancer l'âge de la décote. À ce stade du projet de loi et avant des discussions parlementaires ces ben ces mesures nous paraissent plus équitable que l'allongement de la durée de vie active pour améliorer le taux de pension. Êtes-vous prêt Monsieur le Ministre à corriger ces injustices qui concerne les femmes et que notre groupe a déjà pointé à plusieurs reprises sur un sujet aussi grave. Nous aurons à coeur de trouver en plein dans la majorité sénatoriale, comme à notre habitude, une solution de compromis acceptable par tous, je vous remercie pour votre réponse. Monsieur le ministre du Travail, de l'Emploi et de l'insertion. Je vous donne la parole. Merci monsieur le président, madame la sénatrice Darcos. D'abord vous avez raison sur un point en particulier qui est je crois fondamental dans ce débat sur les retraites et sur les inégalités de niveau de retraite, entre les femmes et les hommes. Aujourd'hui, 50% des femmes retraitées ont une retraite inférieure à 1000 euros brut. Parce que c'est la conséquence l'effet miroir d'une inégalité face au travail d'une égalité face aux salaires et ce mouvement sociologique que nous connaissons d'augmentation du taux d'activité d'augmentation du taux d'emploi des femmes corrige petit à petit et bien trop lentement. Cette inégalité qui est simplement le fruit des inégalités professionnelles et de carrière, c'est là peut-être la priorité, rétablir l'égalité professionnelle pour que nous n'ayons pas au moment des départs à la retraite à imaginer à penser des systèmes de retraite qui soient en réalité des systèmes qui viennent corriger des inégalités accumulés tout au long de la vie. Nous avons dans le projet qui est le nôtre. Un effort qui est demandé à tous les salariés, femmes et hommes, quelle que soit leur cadre d'emploi quel que soit leur camp d'emploi privé public, régimes spéciaux, nous savons que le départ effectif l'âge de départ effectif des femmes va se rapprocher de celui des hommes, même si je l'ai dit tout à l'heure, l'âge moyen de départ des femmes restera inférieur à celui des hommes. Nous avons voulu apporter des corrections et des protections. J'ai évoqué la question de la retraite minimum, vous l'avez fait vous-même je pourrais évoquer par exemple ou révoqué le fait que nous allons intégrer dans les trimestres prise en compte les trimestres cotisés au type de l'assurance vieillesse pour les parents au foyer. Cela concerne 1.900.000 femmes notamment parmi les moins favorisés, tant pour l'éligibilité à la CNAM au minimum de pension que pour l'éligibilité au départ anticipé pour carrière longue. Nous avons certainement encore du travail à faire. Autour de la question des aidants. Nous allons créer cette assurance vieillesse pour les aidants. Ce sont souvent des femmes. Nous avons aussi un travail à faire pour harmoniser les droits. Comment expliquer qu'aujourd'hui une maternité soit génératrices si je puis dire de 4 trimestres de manière automatique otite du régime général et de de au titre de la fonction publique. Nous avons d'ores et déjà demandé avec madame, la Première ministre au conseil d'orientation des retraites d'ouvrir un chantier sur ce sujet-là et j'espère que les débats parlementaires nous permettra d'avancer sur cette question des droits familiaux. Cette question de la parentalité de la maternité mais aussi sur les questions de réversion le texte tel qu'il sera adopté je l'espère, par l'Assemblée nationale nous permettra certainement de construire des consensus. Merci monsieur Ministre j'entends ce que vous dites est en effet. Vous allez déjà revalorisé en effet les plus les plus plus de retraite mais on voudrait pouvoir également parler au nom de toutes ces femmes qui travaillent depuis longtemps, qui ont des, des beaux job et qui ont eu des moments aussi formidable de d'arrêt avec avec leur congé maternité donc de tous les secteurs d'activité, je parle aussi bien évidemment des femmes dans le lieu, l'agriculture, la délégation a fait déjà beaucoup dans d'autres, dans plein de secteur et donc je vous inviterai avec. La secrétaire d'État madame Rome à pouvoir regarder nos nos nos rapports et nos projets pour pouvoir également construire. La fin de ce projet de loi sur les retraites tous ensemble.

Monsieur le président du Sénat, madame, la Première ministre Mesdames et messieurs les Ministres, chers collègues. Il y a un an quasiment jour pour jour paraissait les fossoyeurs. Le livre de Victor Castanet sur le système Orpea. Chacun a salué l'enquête minutieuse et le prix Albert-Londres. Bien méritée. Mais maintenant. Les dysfonctionnements sont connus, les sanctions sont prononcées les EPHAD lucratif doivent être mieux encadrées, puisqu'il prospère du fruit des cotisations et de la solidarité nationale, le Sénat ici a proposé de renforcer le contrôle des Ehpad et si nous avons modifié ce cadre législatif sur le terrain les moyens humains restent lacunaires distant sur pièces comptables, bien loin de nos recommandations pour des inspections contrôle coordonné. Dès lors, les questions subsistent. Monsieur le Ministre de l'autonomie. Entendez-vous nos concitoyennes et nos concitoyens qui espère plus d'attention et de soin pour leurs aînés. Entendez-vous les familles révoltés à juste titre des maltraitances parfois infligés à leurs proches. Entendez-vous l'alerte de la défenseure des droits. Et surtout, Monsieur le Ministre, prenez-vous la mesure de l'attente des soignantes et des soignants qui disent, nous devons être plus nombreuses pour mieux travailler pour cesser de nous a éreintés et pour éviter d'être inapte à l'heure de la retraite. Vous réponde. La parole est au ministre des solidarités. De l'autonomie et des personnes handicapées. Monsieur Jean-Christophe Combe. Merci monsieur le président, mesdames les sénatrices messieurs les sénateurs, madame la sénatrice Michèle Meunier, vous l'avez rappelé il y a un an. Sortait l'enquête approfondie de Victor Castanet, qui a produit une une onde de choc dans notre société, à l'époque j'étais moi-même gestionnaire dans une association gestionnaires d'établissements médico-sociaux et j'ai été profondément choqué par l'ensemble de ces révélations. Depuis lors, je n'ai eu de cesse que de m'engager pour ramener la confiance de nos, de nos concitoyens dans les Ehpad et protéger les personnes âgées, mon rôle aujourd'hui en tant que ministre des solidarités, de l'autonomie et des personnes handicapées, c'est de faire en sorte de poser un cadre de réguler. Un secteur et de faire en sorte que ce cadre soit respecté et je le dis de façon très claire et de façon très ferme. Tous ceux qui aujourd'hui pensent pouvoir se décharger de leur responsabilité en attaquant l'État commettre une double faute. La première, c'est qu'ils mentent aux Français, c'est que, ils ne disent pas la vérité et la seconde c'est qu'à l'époque, ils n'ont pas été à la hauteur et qu'ils ne le sont toujours pas aujourd'hui malheureusement et la vérité c'est que l'État dès les premiers jours de ces révélations, a agi de façon extrêmement puissante en lançant une vague de contrôles inédite avant tous les 20 ans, ces établissements ont été contrôlés, on va les contrôler maintenant tous les deux ans, 1400 établissements sur les 7500 ont d'ores et déjà été contrôlé ont fait l'objet d'inspection, contrôle, grâce au recrutement de 120 contrôleurs supplémentaires dans les ARS et je salue le travail approfondi des ARS pour faire en sorte que ça ne se reproduise pas le 2ème élément que je voulais soulever c'est celui du tabou de la maltraitance contre les personnes adultes vulnérables, il faut lever ce tabou. Libérer la parole je lancerai dans quelques jours, une plateforme de recueil des signalements pour pouvoir libérer cette parole et des états généraux

Madame Meunier. Monsieur le Ministre si vous doutez vous aussi de ce modèle marchand qui ne peut rémunérer des actionnaires que s'il s'occupe mal des personnes âgées. Si c'est le cas, vous trouverez sur nos bancs ici au Sénat des soutiens pourrait mettre fin et ça passera par l'examen d'une loi grand âge elle consacrera cette loi des moyens renforcées et des financements pérennes. Il faut flécher une partie de la richesse créée dans d'autres pays vers la prise en charge des personnes en perte d'autonomie mais les Françaises et les Français ne souhaite pas que cet effort

Donner la parole à notre collègue Valérie Boyer pour le groupe Les Républicains. Merci monsieur le président. Hé oui. Monsieur le ministre, j'associe mon collègue Laurent Somon à ma question. Il y a 3 mois alors que le vice-président du Sénat. Roger Karoutchi vous interroger sur le rapatriement des femmes et des enfants de djihadistes. Vous avez répondu, je vous cite, en réalité notre doctrine n'a pas changé. Ironie ou mépris. En effet, depuis 2009, c'était le cas par cas pour les enfants dans une logique purement humanitaire et la tolérance, 0 pour les femmes et je ne veux employer le terme rapatriement car il s'agit de revenante, nous apprenons par la presse que 15 femmes et 32 enfants sont revenus sans compter les 31 femmes et les 67 enfants l'année dernière. Assumez-vous ce changement de troc Trinh, c'est-à-dire l'abandon du cas par cas et ces retours massifs. Comment. Assurez-vous la prise en charge de ces enfants par les services de l'ASE déjà au bord de l'asphyxie, comme l'enfermement de ces femmes dans nos prisons déjà saturé et qui sont considérés parfois comme des héroïnes, comment pouvez-vous garantir la sécurité des Français face à ces personnes qui haïssent toujours la France.

votre Champ lexical aurait peut être pu vous permettre d'envisager d'autres choses. Nous n'avons pas changé la position du gouvernement est extrêmement claire et elle est précise. Ceux qui ont choisi Daech doivent être jugés au plus près des lieux où ils ont commis leur Crime Mais et ça n'est pas un petit mais. Il y a des enfants madame la sénatrice. Oui, qui n'ont rien choisi et qui doivent être. Traités avec humanité et vigilance. Humanité parce que ce sont des enfants et j'ajoute des enfants français ne vous en déplaise. Et vigilance parce que ils sont susceptibles ment ment susceptible ment possiblement d'être traumatisée à vie avec toutes les séquelles que cela peut engendrer. Alors non, nous n'avons pas changé nous rapatriant à la demande, chaque fois que cela est possible. Des femmes qui le demande, avec des enfants. En ayant naturellement à l'esprit la sécurité de nos forces de l'ordre qui se trouve sur place parce que nous ne maîtrisons pas tout, les femmes ont toutes fait l'objet d'une judiciarisation. Quant aux enfants ils sont placés parfois auprès de leurs grands-parents qui sont des gens parfaitement intégré parfaitement honnête et je le redis parfaitement français, madame la sénatrice. Voilà les enfants font l'objet d'un suivi sanitaire d'un suivi médical d'un suivi psychologique fermeté pour les femmes humanité vigilance pour les enfants on pourrait tomber d'accord là-dessus ça Nelly de l'ironie, ni du mépris. Monsieur le Ministre. L'Humanité vous n'en avez pas le monopole et personne ici ne peut nier que nous aussi nous souhaitons traiter les enfants. En revanche, en revanche. La doctrine du cas par cas avaient été adoptés par vos prédécesseurs monsieur Le Drian et Madame Belloubet. Qu'en est-il aujourd'hui. Pourquoi changer vous de doctrine en opposant désormais pour des migrations mortifère massive. Le président Macron le considéré que ces retours était trop dangereux pour la sécurité des Français. Qu'en est-il aujourd'hui des personnes qui reste combien sont-elles vous injecter dans la population française des djihadistes alors que notre pays est déjà gangrénée par le salafisme. n'oublions pas que la France avec 1400 individus est le 1er pays européen et le 2ème pays au monde à avoir fourni des terroristes à l'état islamiste. Avec des femmes qui se sont engagés pour aller combattre en Syrie et en Irak contre la France. Aujourd'hui, avons-nous les moyens d'une telle politique Les donner la parole à madame la présidente, Valérie Létard. Pour le groupe de l'Union sont. Personne ne peut ignorer ce fléau l'usage détourné du protoxyde d'azote explose en France. Située à la 3ème place des produits psychoactifs, les plus utilisés, notamment chez les jeunes adultes, son caractère addictif est aujourd'hui scientifiquement avéré. Le nombre de cas évalué par les réseaux des centres de pharmacovigilance, qui sont les cas les plus sévères et qui donne souvent lieu à une hospitalisation a été multiplié par 10 en 3 ans. Et ce n'est que la face émergée de l'iceberg, jour après jour, les autorités sanitaires découvrent de nouvelles complications. Suite à cette consommation massive et inédite ces cas. Bien plus grave que d'autres produits qualifiés comme stupéfiant ces cas. Révèle des symptômes psychiatriques anxiété psychose ou autre trouble du comportement. Mais aussi des conséquences lourdes sur la sensibilité la motricité avec des séquelles parfois irréversibles. Pouvant aller jusqu'à une sclérose combinée de la moelle épinière. Face à ce fléau à cette drogue qui ne porte pas son nom. J'ai fait adopter en juin 2021 une première initiative parlementaire pour revenir pour prévenir et encadrer cette consommation détourné avec le soutien de tous nos collègues, Monsieur le Ministre, si je vous interpelle aujourd'hui c'est parce que les décrets d'application de ce texte visant à limiter la quantité de ventes de cartouches de protoxyde mais surtout interdire la vente de bonbonnes à des particuliers devaient être sorti depuis plus de huit mois après avoir alerté votre ministère sur ses retards dès septembre dernier. Il m'a été assuré une publication fin 2022. Pourquoi ces décrets ne sont-ils toujours pas pris quand on sait que les bonbonnes accélère fortement la consommation excessive et régulière de ce, de, Dont les conséquences et son lot de séquelles sont quand même énorme. C'est grave, Monsieur le Ministre. Et d'ailleurs, à quand une véritable campagne d'information et de prévention nationale attendue. Face à ce phénomène toujours croissant et interpellé par les acteurs de terrains professionnels de santé magistrats élus démunis. J'ai déposé un second texte visant à délictuel lisait la consommation de protoxyde d'azote et à poursuivre les personnes qui conduit sur son emprise car c'est extrêmement accidentogène que cela pose un énorme problème. Ministre quand le gouvernement compte se saisir de ce sujet. Président, mesdames, et messieurs les sénateurs, madame la sénatrice les tard je vous rejoins le mésusage du protoxyde d'azote est un problème de santé publique qui touche principalement les plus jeunes, puisque plus de 5 pour des enfants au collège en troisième déclare avoir déjà utilisé ce protoxyde d'azote à des fins récréatives. Alors il y a 2 axes, un axe prévention un axe sanctions comme le le texte que vous avez porté concernant la prévention tout d'abord la connaissance du produit. Vous le dites très bien, on améliore nos connaissances sur ce produit sur sa toxicité. C'est un produit qui est connu depuis longtemps qu'il utilisé en fonction de son pourcentage par rapport à l'oxygène soit comme un gaz anesthésique soit comme un gaz d'antalgiques soi-même comme un gaz hilarant. Ces nouvelles toxicité et que l'on découvre elle touche effectivement le système nerveux central. Mais il ne faut pas oublier une toxicité immédiate en cas d'asphyxie qui est particulièrement dangereuse. L'information est est le fer de lance, nous remontons des informations au niveau national maintenant région par région, ça nous a permis, en particulier dans votre région d'avoir une campagne d'information très ciblée, envers les jeunes entre 15 et 25 en utilisant les réseaux sociaux et nous allons continuer dans cette voie. En ce qui concerne la loi que vous avez porté l'année dernière plusieurs application de cette loi sont déjà en cours, que cela concerne l'interdiction de vente aux mineurs, l'interdiction de vente dans les débits de boisson, l'interdiction de vente des crackers ceux qui sont ces ces dispositifs qui permettent justement ce mésusage tout comme la création d'un délit pour des des personnes majeures qui pousserait des jeunes à l'utiliser en ce qui concerne le la suite de votre projet de loi comme vous le savez cela été notifié à la Commission européenne en février dernier, la commission et le ministère ont fait plusieurs allers-retours un décret, un arrêté sont en cours de publication j'espère avant la fin du mois de février le décret concerne les informations sur les boîtes et sur les produits et arrêté concerne la limitation de vente de 10 capsules maximum par personne. Nous sommes mobilisés face à ce problème de santé publique nous accélérons avec la Commission européenne pour pouvoir publier ses textes au plus vite. Merci la parole est à notre collègue Pierre Cuypers pour le groupe Les Républicains. Monsieur le président, Monsieur le Ministre, je voudrais associer à cette question, la sénatrice Cristina, plus j'ai. Jeudi 19 janvier, jour funeste pour l'agriculture française. La Cour de justice européenne décide de rendre illégales les des des dérogations prévues pour la filière betteravière sur l'utilisation des néonicotinoïdes. Le 30 octobre 2020. Votre prédécesseur affirmait avec justesse que la situation était particulièrement grave et que tout devait être mis en oeuvre pour protéger cette filière. De même, le président de la République affirmer haut et fort qu'il ne devait pas y avoir d'interdit sans solution vous-même Monsieur le Ministre, vous m'affirmiez le 12 janvier être certain de la reconduction de dérogations prévues pour 2023. De plus en 2016, la France a interdit l'usage de tous les néonicotinoïdes en aspersion ou en enrobage de semences, ce que l'Allemagne et tous les autres pays s'autorise. La France s'est mise dans l'impasse. En 2020, la catastrophe de la jaunisse de la betterave avait occasionné 200 millions de pertes. Malgré les engagements pris, l'indemnisation n'a été que de 10 à 30% du préjudice notre souveraineté alimentaire et énergétique et donc menacé, quelles réponses concrètes, le gouvernement entend apporter à cette situation et à cette crise latente. Monsieur le Ministre. Il vous reste moins de 10 jours pour apporter toutes les solutions qui s'impose car les agriculteurs doivent prévoir leurs semis. Pour vous répondre. La parole est oblige d'agricole. Il y aura de souveraineté alimentaire, monsieur Fesneau. Merci monsieur le président, Mesdames, et messieurs les sénateurs, Monsieur le Sénateur Cuypers, vous connaissez très bien cette question et je vous remercie. Avec cette question de pour essayer d'éclairer le débat, vous avez raison, il y a une décision de la Cour de justice de l'Union européenne qui s'impose à tous. Elle vient contrecarrer, disons-le, un plan qui était celui sur 3 ans de sortir des néonicotinoïdes. À la fois en autorisant la dérogation sur les semences enrobées et en permettant de déployer des solutions alternatives et le programme était pour la 3ème année en cours. Cette décision s'impose à nous tous. Vous avez raison, la très peu de temps pour agir pour rassurer les planteurs. Vous l'avez dit aussi d'une certaine forcément pour assurer aussi l'ensemble de la filière. Je pense aux d'industries. Qui triture la betterave et qui sont importantes, en particulier dans votre département dans mes, dans beaucoup de départements de France Première éléments garantir aux agriculteurs qui seront couverts sur la sur la perte de jaunisse, on est en train d'y travailler, mais c'est bien ça sur lequel on doit être au rendez-vous sous les jours qui viennent pour les les assurés qui pourront planté dans des conditions qui soient des conditions d'un d'amortissement, deuxièmement accélérer encore. Les, la recherche de solutions alternatives soit dans celles qui étaient dans le plan national de recherche. Je rappelle qu'on avait mis plus de 20 millions d'euros entre les acteurs de la filière et et l'État, au travers de recherches que mène l'INRA et qu'on travaille avec mes collègues Retailleau et puis 2ème élément d'essayer de travailler sur d'autres recherches et d'autres itinéraires techniques avec des molécules qui sont encore autorisés. J'ai demandé à ce qu'on expertise très vite pour regarder les solutions pour le coin Fowler qui pourrait être expertisé 3ème élément. Vous avez raison, Monsieur le Sénateur, je maintiens ce que a dit mon prédécesseur, ce qu'a dit le président de la république et ce que j'ai dit pas l'interdiction sans solution. La vérité c'est que cette interdiction et le procès de 2016. Le principe de précaution à la charte de l'environnement et des il date de bien avant donc c'est il faut qu'on assume aussi les décisions qui ont été prises. C'est difficile pour tout le monde y compris pour le ministre de l'Agriculture. C'est difficile, surtout pour les betteraviers. Moi, mon sujet, c'est de leur donner de la visibilité, la visibilité, c'est le plan de soutien sur la jaunisse et c'est de d'associer aussi les transformateurs, pour faire en sorte que il se dit il bénéficie des betteraves dont ils ont besoin pour faire tourner les outils de production. Nous allons-y travailler dans les jours qui viennent, nous nous sommes déjà à l'oeuvre. Je connaissais votre réponse. Mais il faut des solutions et des certitudes parce qu'au-delà de la compréhension. Au-delà de l'impuissance française c'est la colère, c'est le désarroi. C'est le feu dans nos territoires c'est le saccage annoncé de nos filières, c'est la mise en péril de l'industrie du sucre, de l'alcool du bioéthanol du gel hydro-alcoolique de l'alimentation animale, ça ne risque d'importation massive de ce coup d'éthanol notamment du Brésil, qui est produit avec des produits que nous refusons ici en France cette obéir là c'est obérer la souveraineté alimentaire et énergétique, la France Cook devient le seul pays au monde à tous ces interdits.

Madame, la Première Ministre Mesdames messieurs les gouvernements, mesdames, messieurs, chers collègues. Ma question s'adresse au ministre de l'Intérieur. Cela fait 4 mois que l'Iran connaît un mouvement citoyen inédit afin de dénoncer le régime théocratique ces violations des droits fondamentaux et des libertés publiques. Comme vous le savez, ce mouvement est né au lendemain de la mort de. Mahsa Amini, accusé de ne pas avoir porté correctement son voile. Depuis, ce sont surtout des femmes et des hommes qui sont à la pointe de cette mobilisation. En retour, la répression du régime est implacable. Des milliers d'arrestations, 500 morts des simulacres de procès, les exécutions sommaires. Persécuté par le régime iranien des opposants fuit l'Iran et trouve refuge pour certains en France. C'est le cas de Farideh une iranien de 38 ans interpellé la semaine dernière par la police aux frontières à l'aéroport de Chambéry, alors qu'elle souhaitait se rendre en Angleterre pour rejoindre son mari. Là-bas. Elle fut ensuite transféré au centre de rétention administrative de Toulouse enfermé pendant 48 heures avant d'être libéré. Pendant que la préfecture prenait une obligation de quitter le territoire français et contacter les services consulaires iranien en France afin d'envisager sa reconduite à la frontière, comme c'est le cas et comme c'est l'usage à chaque fois qu'une obligation de quitter le territoire est prise. Cela nous interpelle. Soit nous interrogent parce que la France, à l'instar des autres pays occidentaux, par la voix du président de la République de plusieurs ministres ici présents à condamner la répression en oeuvre en Iran et apporté son soutien aux manifestants. Monsieur le ministre de l'Intérieur, pouvez-vous nous préciser la doctrine de la France à l'égard des opposants au régime iranien présent notre pays qu'ils soient en situation régulière ou irrégulière. Pour vous. Car monsieur le ministre de l'Intérieur. Les deux premières monsieur Darmanin. Merci monsieur le président, Mesdames, et messieurs les sénateurs, monsieur le sénateur. La citoyenne iranienne que vous évoquez, a été interpellé 4 fois sur le sol national et lors de sa première interpellation lorsque les services de la police aux constaté qu'elle était pas régulièrement sur le territoire national et qu'elle se disait tu iranienne. Il fallait évidemment vérifier son identité. Et c'est pour cela que nous consultons les services consulaires de tous les pays, c'est le cas évidemment pour l'Iran avec qui nous avons encore des relations diplomatiques pour identifier des personnes afin qu'elle ne se fasse pas passer pour une autre personne. Une fois que nous avons constaté en effet qui était iranienne. Nous l'avons libéré comme vous l'avez très bien dit du centre de rétention. C'est l'État qui l'a fait et ce n'est pas un jugement administratif. Vous avez oublié de le mettre. Vous avez oublié, pardon de le lire. Et deuxièmement, nous lui avons encouragé, nous l'avons encouragé à prendre des rendez vous pour pouvoir demander l'asile dans notre pays ou un titre de séjour afin de régulariser sa situation. Elle ne l'a jamais fait. Après ce 1er contrôle trois autres contrôles ont été constatés par la police aux frontières. La République ne peut pas accepter quelqu'un qui est irrégulièrement sur le territoire national. Cette personne ne veut pas rester en France, elle ne veut pas demander l'asile en France. Elle ne veut pas de titre de séjour en France, nous l'aurions accueilli évidemment mais elle veut rejoindre comme vous l'avez dit, sa famille qui est en Angleterre. Il ne s'agit donc pas pour la France de ramener vers l'Iran des ressortissants nous ne ramenons pu évidemment vers l'Iran des ressortissants nous identifions les personnes s'ils ne veulent pas rester sur notre sol. On va pas leur donner des papiers de force avouez bien volontiers les choses et nous avons contacté le Royaume-Uni pour qu'elle puisse se rapprocher de sa famille. Nous n'avons pas encore reçu. Réponse de la part du gouvernement britannique. Mais je veux ici vous assurer que des seront personne et encore moins la personne que vous évoquez en Iran. Nous le réinvite ont et si vous avez contact avec elle. Je vous demande de le faire si elles le souhaitent, de déposer un dossier demande d'asile en France, nous l'étudierons évidemment avec rapidité et avec humanité. Monsieur le Ministre, je vous remercie pour la réponse. Mais comme vous le savez, son mari est en Angleterre c'est là-bas qu'elle compte faire ces démarches. Je voulais vous dire Monsieur le Ministre, que l'histoire de notre pays. Elle est grande, elle est belle, elle nous donne chaque jour à chacun à chacune d'entre nous, des motifs légitimes d'en tirer une fierté particulière. Parfois, elle connaît des zones d'ombres. Cette histoire de France. Lorsque nous n'avons pas su ou pas voulu apporter la protection nécessaire à ceux qui travaillaient pour l'armée française en Afghanistan, les fixeurs, les grilles, les traducteurs. Je vous demande, monsieur le ministre et je m'adresse à vous en tant que ministre et je m'adresse surtout à votre conscience à veiller à ce que les 50 iraniens qui sont aujourd'hui sous le coup d'une OQTF ne soient pas renvoyés dans leur pays, car vous connaissez très bien le sort qui pourrait leur être réservé, je parle de cette dame mais je parle de coupures faute La parole est à notre collègue Olivier Paccaud pour le groupe Les Républicains. Merci monsieur le président. Ma question s'adresse au ministre de l'Éducation nationale, Monsieur le Ministre, dans le calendrier révolutionnaire. Nous sommes en pluvieuse c'est le mois de la pluie et il pleut des annonces de fermetures de classes partout dans le pays, surtout en zone rurale.

indispensable des rémunérations des enseignants. Mais alors que tous les classements internationaux toutes les. Évaluations nationales, alerte sur la fragilisation de du niveau global des élèves, alors que vous vanter les vertus, les effectifs réduits et des classes dédoublées. Où est la cohérence pédagogique et surtout où est la justice territoriale quant à quelques km quelques hectomètres parfois ici on va fermer une classe parce qu'avec 22 gamins ils sont trop nombreux et à côté on va se réjouir d'avoir 12 gamins dans une classe dédoublées pour plus d'efficacité, je le rappelle, 70% des élèves qui relève de l'éducation prioritaire, se trouve en zone rurale ou dans des quartiers qui ne sont pas concernés. Monsieur le Ministre, ma question elle est simple, la ruralité est-elle devenue la variable d'ajustement de vos politique éducative.

Merci monsieur le président, Mesdames, et messieurs les sénateurs, Monsieur le Sénateur Paco, vous l'avez dit la. Démographie scolaire connaît une baisse importante depuis plusieurs années une baisse qui va s'accentuer au rythme de 90.000 à 100.000 élèves de moins chaque année, nous prévoyons une baisse donc de d'environ 500.000 élèves d'ici. À la fin du quinquennat dans votre département de l'Oise par exemple ce sont 1367 élèves que l'on va compter en moins à la prochaine rentrée. Dans ce contexte de baisse démographique, le taux d'encadrement, c'est-à-dire le ratio entre professeurs et élèves s'améliore depuis plusieurs années, il va continuer à s'améliorer, par exemple dans l'Oise. Il y a en moyenne 21,5 pour 21,5 élèves par classe et cette moyenne va s'améliorer légèrement l'année prochaine nous avons créé ces dernières années sans de postes de professeurs dans l'Oise pour une baisse de 6631 élèves dans le budget 2023, nous avons, comme vous l'avez dit, donner la priorité à la revalorisation des professeurs parce que monsieur le sénateur, à quoi sert-il de créer des postes, si nous ne pouvons pas pourvoir les postes. La question est donc d'abord de pourvoir les postes que nous créons avant de les multiplier sans que cela ait un effet sur le terrain. Quant aux fermetures que vous évoquez, nous ne le faisons pas de manière arithmétique, bien au contraire dans chaque département les Dasen sont au je suis particulièrement sensible moi même à la situation des zones rurales et des écoles rurales de manière à faire des ajustements en juin et en juin et également en. En août, à la fin août. À ce stade rien n'est définitivement arrêté et je serais heureux d'en reparler avec. Évoquer la ruralité parce que un des gros problèmes de l'Éducation nationale, mais même des politiques publiques depuis des années, c'est l'oubli de ses territoires en 19 47, Jean-François Gravier publié Paris et le désert français depuis 2017. Emmanuel Macron décline les métropoles et le désert français, la France c'est 101 départements, 35.000 communes, 68 millions d'habitants et la République, c'est aussi et surtout l'égalité des droits et des chances partout et pour tous.

Je m'adresse à tous les ministres tant le sujet nous concerne tous. Savez-vous que la présidente de la Commission européenne a autorisé le 3 janvier dernier un nouvel aliment. Savez-vous que ce nouvel aliment est une farine partiellement dégraissé incorporé dans de multiples recettes. Savez-vous que depuis hier vous pouvez trouver cette farine sans information claire du consommateur dans les pins biscuits, sauces plats transformés pizza confiserie ou pâte et j'en passe et des meilleures. Enfin, savez-vous que cette farine partiellement dégraissé et fait avec des acheta domestique us entiers broyés en poudre.

Merci monsieur le président, Mesdames, et messieurs les sénateurs. Oui, monsieur le sénateur, je crois que c'est un insecte. Et donc c'est bien la question. Vous voulez poser c'est de savoir d'abord pour dire que. Pardon de vous le dire, il n'est pas nouveau, y compris dedans depuis très longtemps que dans un certain nombre de pays on puisse se nourrir d'insectes. Ça n'est pas en soi, on peut avoir des goûts différents, moi compris. Mais c'est une réalité 2ème élément ça participe tout à fait d'une réglementation européenne qui a été autorisé simplement la réglementation européenne exige. Monsieur le sénateur, c'est qu'on mentionne. La nature du produit, en l'occurrence pour ce, ce, cet insecte la caisse. La question de l'allergénicité. Des uns et des autres, donc il faut qu'on soit vigilant sur la mention dans les produits qui seront dans disant ans qu'il a un produit qui peuvent être allergènes en l'occurrence cet insecte 3ème élément au travail au niveau européen globalement essayer d'harmoniser les choses et c'est mieux que ça soit au niveau européen que chaque pays décide. De commercialiser telle ou telle autre et donc c'est ça sur lequel on a besoin de travailler, ça nécessite aussi et nous avons besoin de continuer à renforcer à nos frontières européennes mais aussi au niveau national la surveillance sanitaire parce qu'il y a toujours des gens qui essaient de déroger aux règles que nous nous fixons au niveau européen. Ça existe dans le sujet agricole et sanitaire, comme dans bien d'autres sujets. Donc il faut qu'on y travaille, qu'on continue à avancer mais reconnaissons que les mesures qui sont prises elles vise plutôt à protéger à informer le consommateur à protéger le cas échéant, l'environnement et donc c'est là dessus qu'il faut qu'on travaille sans travailler sur des questions distorsion de concurrence un permis de. Un dernier mot monsieur le sénateur. Ils sont que sur ces sujets, il faut qu'on le travaille justement au niveau européen. Rien ne s'est pris, on en a parlé dans un autre exemple, tout à l'heure que d'avoir des dispositions qui s'applique simplement sur le sol français qui ne s'applique pas au niveau européen, donc la bataille, elle est d'abord européenne et c'est là-dessus qu'il faut qu'on continue à travailler. Monsieur le Ministre, comment en sommes-nous arrivés là. À devoir consommer des grillons. De la même famille que les sauterelles ou les criquets, alors que la France est le pays de la gastronomie et des terroirs. Comment pouvez-vous laisser faire cela alors que vous n'avez de cesse de nous parler d'une alimentation saine et durable d'agroécologie et de circuits courts saine et durable, cette farine ne l'est pas. Même la Commission ne garantit pas l'absence de problème sanitaire. Contrairement à ce que vous venez de dire, où est l'agroécologie. Avec l'élevage hors sol de millions de grillons dans des bâtiments industriels. Et que dire des circuits courts, alors que cette poudre de grillons est importé du Vietnam. Cette commission européenne qui cède aux lobbies anti-viande et qui sape notre agriculture et notre culture gastronomique. Je n'en veux plus soutenant plutôt la farine de blé française plutôt que la farine de grillons soutenant le suc aux Français plutôt que les insectes d'Asir. Nous ne pouvons pas accepter de faire manger à leur insu des insectes aux Français qu'qui souhaitent manger des grillons, Monsieur le Ministre, je les invite à venir les manger directement dans mes. Ils sauront nature entier non broyés et non transformés et pour tous les autres, je leur conseille de constituer que de continuer à manger une bonne côte de boeuf. Mes chers collègues. Après ses recommandations gastronomique. Je vous rappelle. Et là c'est un une annonce particulièrement importante que mercredi 1er février à 14h 30 nous recevrons monsieur Rouslan Stefantchouk, président de la Rada d'Ukraine dans notre hémicycle et qui s'exprimera. Je compte particulièrement sur la présence de chacune et de chacun. D'accord avec le gouvernement, les questions d'actualité débuteront donc à titre exceptionnel avec 15 minutes de décalage donc à 15h 15. Je vais maintenant suspende la séance sera reprise. À 16h 30 pour l'examen de 3 conventions internationales puis pour la suite de l'examen du projet de loi relatif aux Jeux olympiques et paralympiques de 2024. La séance est suspendue.

La commission des finances a émis lors de sa réunion de ce jour un avis favorable. 19 voix pour aucune voix contre. À la nomination de Monsieur Robert Ophèle à la présidence de l'Autorité des normes comptables. L'ordre du jour appelle l'examen de 3 projets de loi près tendant à autoriser la ratification l'approbation de conventions internationales pour ces 3 projets de loi, la conférence de présider président a retenu la procédure d'examen simplifiée. Je vais donc les maîtres successivement aux voix. Je mets aux voix donc pour commencer le texte adopté par la commission sur le projet de loi autorisant l'approbation de l'amendement de la Convention relative à la collecte au dépôt. Et à la réception des déchets survenant en navigation rhénane et intérieure et de son règlement d'application. La commission des Affaires étrangères de la Défense et des forces armées et favorable à l'adoption de ce texte. Qui est pour. Qui est contre. Le projet de loi est adopté, je mets aux voix. Le texte adopté par la commission sur le projet de loi adopté par son. L'Assemblée nationale après engagement de la procédure accélérée, autorisant l'approbation de l'accord entre le gouvernement de la République française et le gouvernement du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord, relatif à la coopération sur les questions de sûreté maritime et portuaire. S'agissant spécifiquement des navires à passagers dans la Manche. La commission des Affaires étrangères de la Défense et des forces armées et favorable à l'adoption de ce texte qui est pour. Qui est contre. Qui s'abstient. Le projet de loi est adopté définitivement, je me vois le texte adopté par la commission sur le projet de loi adopté par l'Assemblée nationale, autorisant la la l'approbation de l'accord entre le gouvernement de la République française. Et le gouvernement de la République d'Ouzbékistan relatif aux transports routiers internationaux de voyageurs et de marchandises. Et de l'accord entre le gouvernement de la République française. Et le gouvernement de la République tunisienne sur le transport international routier de personnes. La commission des Affaires étrangères est favorable à l'adoption de ce texte qui est pour. Qui est contre qui s'abstient. Le projet est adopté définitivement. L'ordre du jour appelle la suite de l'examen du projet de loi relatif aux Jeux olympiques et paralympiques de 2024. Dans la discussion des articles. Nous sommes parvenus à l'article 13. Et concernant l'article 13 je passe la parole à monsieur dessus pour un amendement l'amendement numéro 69. Merci, monsieur le Président Madame la Ministre donc on arrive sur l'article 13 qui concerne les interdictions judiciaires de stade qui pour nous n'ont pas grand rapport avec les Jeux olympiques. Alors on a beaucoup parlé hier. Du des événements du Stade de France et du rapport et des auditions qu'on a pu avoir. Au Sénat, et parmi les recommandations qui ont été. Émises. Par ce rapport, il y en a une qui bizarrement n'a pas retenu l'attention. De la ministre ou du ministre de l'Intérieur, je parle de la recommandation numéro 13 qui, dans un souci de faire disparaître comme nous le souhaitons tous La violence dans les stades préconisait je cite de faire évoluer le regard des autorités publiques sur les supporters et créer les conditions d'un dialogue permanent, afin de faire de leurs représentants des partenaires dans le cadre de la préparation et du déroulé des grands événements. supporters et les associations de supporters a été consulté pour cet article, puisque. Comme à son habitude, le Sénat a préféré la répression la répression rien que la répression, puisque le Sénat comment comme à son habitude ne presque ne prêche pas pour le dialogue, mais pour le Tour de vices répressif rends les interdictions de stade obligatoire pour un certain nombre d'infractions est une mesure aussi disproportionnée qu'aberrante dans le cadre d'un projet de loi sur les jeux olympiques. Nous sommes encore ici sur un article qui. Se sert des Jeux olympiques comme d'un prétexte, Quel rapport entre les épreuves de gymnastique et les interdictions de stade que si à ce que ce qu'on est-ce qu'une si une personne perturbe une compétition de gymnastique lors des JO. Est-ce que se verra interdire est obligé de pointer les soirs de compétition nationale de gymnastique au commissariat je vous voulez bien que tout ceci est absurde a concerne effectivement les compétitions de football mais pas les JO donc toujours dans notre logique de distinguer si concerne les jeux et ce qui va au-delà. Nous vous proposons de rejeter de supprimer cet article. Merci. L'avis de la commission. Merci, monsieur le Président Madame la Ministre. Mes chers collègues. Contrairement à ce qu'indique l'objet de cet amendement les les intrusions sur les aires de compétition visés par le nouvel article L hein ne sont pas concernés par la nouvelle interdiction obligatoire de stade créé par l'article 13, ces indus intrusion relèveront d'une interdiction facultative, dont on sait qu'elles sont très rarement prononcées par les juges les entre les interdictions obligatoire viseront uniquement les délits les plus graves commis dans les enceintes sportives. C'est donc un avis défavorable. Monsieur le sénateur dessus. Monsieur le rapporteur. Également un avis défavorable sur ce sur ce point. Pour les mêmes raisons. Je voudrais vraiment souligner que ces interdictions judiciaires de stade précisément en consultant l'ensemble des 47 membres de l'instit de l'instance nationale du supportérisme. Les principales associations de supporters. Nous avons recentré la systématisation de ces interdictions judiciaires de stade aux seules infractions délits les plus graves. Donc l'introduction dans un stade objet susceptible de constituer une arme l'incitation à la haine, l'incitation à la violence. L'invitation aux discriminations. Ce sont ces 4 éléments je rappelle d'autre part que c'est une mesure prononcée par le juge qui conserve la faculté de ne pas prononcer cette interdiction judiciaire de stade. Merci donc un double avis défavorable. Pas de demande d'explications de vote, je. Allez-y monsieur Bruno. Merci monsieur le président. Moi je, je suis très intéressé par ce débat malgré tout parce qu'on a dit que c'était une une mesure visant notamment dernière génération.

Sur ces soi-disant militants qui au nom de motif supposé manque de connaissance de préservation de la planète, viennent perturber les opérations sportives les manifestants sportive comme ça, c'est vous à Roland Garros et qui, non content de bloquer parfois les routes et et de de flûte de flux des personnes qui travaillent à 8h du matin comme ça s'est passé sur certaines périphérique avec des, des menaces et des violences. Pour le coup, dont ils sont responsables, qui donc ils ne répondent pas toujours. Je voudrais quand même voulu m'administrer que vous ayez un mot particulier par rapport à à ce type de de militants qui, au motif de protéger la planète, viennent non seulement perturber les manifestations mais mettre en danger la vie d'autrui. Hier nous parlions d'autre chose et nous parlions effectivement de militants qui, pour avoir une audience utilise un certain nombre d'événements sportifs pour pouvoir montrer et faire

par les manifestations violentes qui peuvent exister ici ou là. Oui je suis d'accord il y a il y a même les défenseurs de la chasse ou de la propriété privée qui peuvent bloquer les autoroutes et les routes qui peuvent bloquer les péages c'est Viola et pour autant. Voilà je dis. Mais pas tous dans le même palier donc s'il vous plaît chers collègues soyons de soyons pas manichéens. Voilà soyons calme rien de doux presse de légiférer là c'est tout à fait autre chose. La question que posait monsieur Dossus c'est tout simplement à partir du moment où on voit à supporters

s'il y a une compétition aux Jeux olympiques de gymnastique rythmique et qui a un supporteur violents qui vit à intervenir en valent condamné à quoi administrativement en fait a pu assister à une compétition de gymnastique sportive lorsqu'on en a discuté avec le ministère. On m'a dit oui mais si les supporters de clubs s'il est inscrit dans un club, on va essayer d'aller chercher dans quel club il est comment. Pour le punir et pour l'obliger. Avec une sanction administrative à 2 pas assister à des compétitions de son club etc tout ça nous paraît pas du tout opérationnel dans la réalité et en plus à ce que le public des JO c'est le public justement qu'il va falloir cibler avec ces mesures là où est-ce que c'est une mesure qui est faite pour après les JO, comme beaucoup d'autres dans le texte si juste là-dessus quand vous les bateaux Focus. Merci madame la ministre. Monsieur le président. Je voulais juste. Réagir pour dire que ce qu'Alain a bien été couvert hier avec l'adoption de l'article 12 qui crée un nouveau délit. pour introduction sur une aire de jeux sans motif légitime, là on est dans cet article 13 sur cet enjeu des interdictions judiciaires de stade dont la dimension de pointage est au coeur. De la vocation dissuasive. Merci donc je vais soumettre aux voix. Cet amendement de suppression qui est pour. Qui est contre. Qui s'abstient. Il n'est pas adopté l'amendement suivant le 85. Choubaki. Merci, monsieur le Président Madame la Ministre, mes chers collègues. Il nous semble nécessaire de remplacer le terme obligatoire par celui d'automatique, c'est pas qu'une bataille sémantique en effet tandis que l'obligation renvoie un mécanisme de contraintes et semble restreindre toute possibilité de dérogation motivée à l'appréciation du tribunal l'automaticité renvoie quant à elle, davantage à une logique de présomption. L'usage du terme d'automaticité nous semble ainsi plus cohérent et permet de donner davantage de pouvoir d'appréciation au tribunal. Par ailleurs, il nous semble aussi au Porto ne prévoir que l'absence de risque de récidive doit être prise en compte pour décider d'une dispense d'IDS je vous remercie. Merci monsieur le président, madame la ministre, chers collègues. Mon chérie, mon collègue là qui. C'est vrai que cet amendement prend propose de rendre automatique plutôt. Qu'obligatoire les interdictions de stade pour les délits les plus graves. Je peux comprendre la démarche. Malheureusement, il faut savoir que l'automatiser l'. Automaticité pardon d'une peine reviendrait à remettre en cause le principe constitutionnel de l'individualisation des peines. La rédaction actuelle prévoit ainsi que le juge pourra décider par une décision spécialement motivée de ne pas prononcer cette peine. C'est donc un avis défavorable. Monsieur le président. Même avis dans la mesure où ce terme cet adjectif d'obligatoire hé bien celui que l'on retrouve dans notre. Dans et introduire cette idée d'automaticité ne permettrait pas de rendre compte du fait que le juge peut en effet spécialement de manière spécialement motivée décider de ne pas prononcer cette IGS donc dire automatique donnerait l'impression qu'on abdique le jugement. Le sens du jugement et donc. C'est moins adapté. Donc un double avis défavorable ou le retirer, il est retiré l'amendement suivant le 83 Monsieur Merci, monsieur le Président Madame la Ministre. Les supporters partout dans le monde utilisent des torches et des fumigènes pour animer les tribunes leur interdiction n'empêche pas la pratique de perdurer et sa répression conduit à rendre leur utilisation encore plus dangereux. En effet, pour contrer cette interdiction lors des fouilles certains supporters de plus en plus nombreux, on peut le regretter, réduisent la taille des engins pyrotechniques ancien notamment les partis qui permettent de protéger les mains de l'utilisateur en août pour éviter d'être reconnu au moment d'allumer et donc d'allumer les bras tendus devant eux, les engins sont allumées, sous des bâches non ignifugée des ainsi les risques. Un rapport parlementaire de mai 2020, souligne d'ailleurs que la dangerosité des fumigènes étaient imputable notamment leur interdiction. Par ailleurs, la répression est totalement inefficace Rendez-vous compte dans quelques années nous sommes passés de quelques centaines à plusieurs milliers d'engins pyrotechniques utilisés par conséquent. Force est de constater que l'interdiction qu'inapplicables. Vouloir la renforcer davantage et tout bonnement hypocrite, selon nous, de plus elle engorge les tribunaux devant traiter de aussi dérisoire comme un délit. Et en fait elle m'apparaît irresponsable pour les raisons en matière de sécurité, que j'évoquais précédemment. En revanche, l'usage d'objets d'étonnant je pense au pétard aux bombes agricoles ou autres, ou l'utilisation d'une torche comme projectiles ou armes ne participe nullement à l'animation des tribunes et sont à l'origine des blessures constatées lors de certaines manifestations sportives et ils doivent donc rester formellement interdit et lourdement sanctionné, je vous remercie. Merci, monsieur le Président Madame la Ministre, mes chers collègues. L'article L. 332 tiré 8 du code du sport prévoit que le fait d'introduire des fusées ou artifices sans autorisation dans une enceinte sportive est puni de 3 ans de prison et de 15.000 euros d'amende avec. Ce présent amendement pardon vise à supprimer cette peine de prison et à ramener l'amende à 150 euros. Je m'interroge sur le choix retenu soit le fait d'introduire ces fusées sans autorisation dans une enceinte sportive ne pose pas de problème et il convient de l'autoriser ou de supprimer toute sanction soit on considère que l'absence d'autorisation de règles d'emploi et de contrôle sur l'origine et et la sécurité de ces engins. Pyrotechniques et susceptibles de porter atteinte à la sécurité des spectateurs et dans ce cas il ne, il convient de ne pas modifier le droit en vigueur. Sans être opposé par principe à l'à l'usage de ces engins lorsque celui-ci est encadrée. Et contrôlée par les organisateurs. Je ne peux qu'être défavorable à ce qu'un usage anarchique ne soient plus sanctionnés, alors que la sécurité dans les stades est redevenu un sujet préoccupant. Même avis défavorable. Je voudrais souligner un point, vous, vous avez en tête que ce délit a été créé en 92 et que dans la loi du 2 mars 2022. On a prévu une expérimentation encadré de la pyrotechnie, qui fait l'objet d'un décret qui sera prêt un décret en Conseil d'État qui sera prêt fin mars qui a été soumis aux associations de supporters et qui nous permettra d'aller au bout d'une expérimentation pour une démarche de pour une durée de 3 ans, au terme de laquelle il faudra en effet que nous tirions toutes les conclusions avec les associations de supporters avec les forces de sécurité de l'usage de qui aura été fait de cette pyrotechnie pour vraiment la prendre cette décision de demeurer au niveau du délit ou bien de convertir enfin on une contravention. Merci monsieur le rapporteur. Merci madame la ministre. L'objet de cet amendement, c'est aussi de pouvoir réparer je dirais une certaine hypocrisie ce selon moi l'hypocrisie consiste à dire que ces engins sont interdits dans nos stades parce que potentiellement dangereux. Mais dans le même temps vous avez des spots publicitaires de ligues sportives. Vous avez des spots publicitaires de diffuseurs qui utilise toutes ces images de stade avec des fumigènes, les engins pyrotechniques parce que ça participe à l'idée d'un sport populaire très large. La passion et cetera donc moi ce que je demande c'est qu'on puisse mettre en adéquation, en réalité, ce qui est promue par un certain nombre d'instances dans ce pays avec la législation. Je sais bien qu'il y a effectivement. Pour le coup une expérimentation qui a été mis en place, je sais que des clubs comme Toulouse par exemple auront pu en bénéficier jusqu'à présent on ira au terme évidemment, mais jusqu'à présent du sang des choses semble plutôt bien se passer. je j'appelle à corriger justement cette hypocrisie. Même si j'entends vos arguments. Je vous remercie. Merci. Donc je vais soumettre aux voix cet, cet amendement le 83 avec un double avis défavorable qui est pour.

Ce projet de loi rappelle à son article 13 que l'interdiction judiciaire de stade et l'interdiction de principe. Par conséquent, il convient de préserver les libertés fondamentales et l'État de droit en ramenant les traditions administratives à sa plus juste mesures préalables, force est de constater les nombreuses et graves dérives dans l'application de ces mesures de police administrative fortement attentatoire aux libertés fondamentales, il est préconisé de revenir à une durée plus proche de celle prévue. Par le législateur qui était de 3 mois d'ailleurs le rapport parlementaire de mai 2020 souligné je cite la surenchère continue entre 2006 et 2016, qui a conduit à multiplier par 12 la durée des IAS Plus loin, le rapport préconisait de fixer la durée maximale des IS à six mois et à 12 en cas de récidive. Je profite de ce temps de parole pour rappeler à quel point il est fondamental de garder en tête que les mesures de police administrative sont des mesures d'urgence prises en attendant que l'autorité judiciaire, n'engage une procédure il ne prononce une interdiction de stade de telles mesures ne saurait constituer des sanctions prises durablement seule l'autorité judiciaire est à même de prendre des mesures privatives de liberté dans le temps, je vous remercie. Merci, monsieur le Président Madame la Ministre, mes chers collègues. Cet amendement vise à réduire drastiquement la durée maximale de l'arrêté portant interdiction de stade. Les interdictions de stade étant particulièrement dissuasive. Cet amendement aurait pour effet de réduire qu'on s'est considérablement l'arsenal juridique permettant de lutter contre les contre les violences dans les stades alors que ces phénomènes ont plutôt tendance à se développer. Depuis la fin de la crise sanitaire. Donc une ah en ce moment une telle évolution n'apparaît ni opportune ni souhaitable. Alors que nous avons de manifestations sportives majeures qui sont attendus en France en 2023 et 2024. Donc, avis défavorable. Merci, madame la Ministre votre avis. Durée de 2 ans, maximum trois ans étant le maximum mais le préfet prouvant toujours décidé une durée moindre. Merci donc je vais soumettre. Monsieur j'ai juste une question parce que j'ai été interpellé un peu par la réponse du du. Du rapporteur. Pour bien comprendre, les chiffres que dans nos pouvoir disposer fait si j'ai bien compris on on sait que c'est pas une sont dissuasive. Mais en même temps, c'est que le phénomène augmente. Donc en fait je me posais la question de savoir si qu'elle était la relation entre les deux, donc autrement dit, ça veut dire que si il n'y avait pas ces peines dissuasif le phénomène augmenterait encore plus. Est ce qu'on a des éléments qui nous permettent de de passer ça à ce qu'il y a des éléments chiffrés à ce qu'on sait quel est l'impact réellement de ces pannes augmenter veut c'est un peu ma question, ça m'est venu. Bien je vais soumettre aux voix cet amendement avec un double avis défavorable qui est pour cet amendement.

La mesure de pointage au commissariat à chaque rencontre est excessivement lourde pour bon nombre de nos concitoyens pour supporter d'un club qui joue plusieurs compétitions elle peut le comprennent à se rendre au commissariat jusqu'à 70 fois dans l'année, au détriment de sa vie personnelle social professionnel familiale ou associative. Cette procédure est également démesurément contraignante lorsque le justiciable cherche à obtenir de la préfecture l'autorisation de partir en week-end en vacances ou en déplacement professionnel, la plupart du temps les préfectures ne répondent pas ou refusent ce qui oblige les supporters à saisir les tribunaux administratifs et le Conseil d'État en référé en août. Certaines préfectures en abus sans en mesurer la conséquence concrète dans la vie de certains supporters ici, je pense par exemple à la préfecture de police de Paris ou encore. À la préfecture du Pas-de-Calais qui ont visé un si grand nombre de manifestations sportives que les supporters devraient Ponté pointé 15 fois par semaine. Ici encore, la saisine du juge administratif en référé fut nécessaire pour corriger ces dérives pourtant la mesure de pointage n'a pas vocation à être automatique. Cette mesure ne peut se justifier que si elle apparaît strictement nécessaire pour prévenir un risque de trouble grave à l'ordre public, tel est le sens de notre amendement d'autant plus qu'il existe déjà à l'article L.. 332 tiré 16 qui vise à dissuader un supporter de méconnaître une interdiction administrative de stade hein prévoyant un an d'emprisonnement d'emprisonnement et 3750 euros d'amende pour celui ou celle qui ne se conformera pas à l'arrêté de la préfecture. En fait, il est apparu dans la pratique, une telle généralisation de l'obligation de pointage engendre un fort encombrement des commissariats ou des gendarmeries à des horaires où ils sont déjà malheureusement en sous-. Effectif. Je vous remercie. merci Monsieur le Président Madame la Ministre, mes chers collègues. Cet amendement vise à supprimer donc l'obligation de pointage pour les interdits de stade, alors que cette. Obligation est particulièrement dissuasive et efficace. ne mais c'est mésestime pas la difficulté d'application de cette disposition. Même si ces interdictions de stade ne sont pas aussi nombreuses que cela pourrait être des fois nécessaire. en réponse également à monsieur Bena Roche. Nous avons oh no au nom de la commission. Adopté un amendement à l'article 13 qui enjoint le ministère de l'Intérieur nous fournir des données sur les violations des interdictions de stade. Dans l'immédiat, il apparaît donc inopportun d'affaiblir un dispositif particulièrement utile pour lutter contre la violence dans les stades, donc c'est un avis défavorable. Oui. Avis défavorable également parce que c'est une mesure qui était efficace qui est utile et qui est dissuasive. Comme nous l'avons dit précédemment, le préfet a toujours. La faculté de ne pas renoncer, ça et, en outre, dans ces mesures là on a une logique de protection aussi des droits des personnes avec une obligation de motivation le contradictoire la proportionnalité donc un ensemble de garanties qui sont également. Non négligeable dans notre droit.

L'article 12 et et l'article 13, c'est-à-dire ce qui concerne le durcissement des peines. Initiée par par le Sénat cette ce durcissement des peines concernent essentiellement l'article 12 et non pas l'article 13, un article donc nous avons examiné hier mais ce que je voulais dire en ce qui concerne notre état d'esprit à nous c'est que globalement. Je dirais que les positions qui avait été transmise communiqué par le gouvernement, par le Conseil des ministres et nous paraissait plutôt satisfaisante. Dès lors que l'avis de la CNIL est l'avis du Conseil d'État était étaient prise en compte mais ce que je voudrais ajouter, c'est que notre notre vigilance va va se poursuivre au cours des des mois et même des années qui viennent parce que cet article 13, c'est l'illustration même. D'un texte qui n'est pas simplement un test olympique mais également un test post-olympique. Puisqu'il y a effectivement des une concertation qui est en cours. Des discussions qui se poursuivent notamment des discussions inter-. Ministérielles mais également avec les instances qui représente les supporters et donc probablement je pense à un certain moment, toutes ces discussions-là auront un débouché politique à travers un texte de loi qui viendra prolonger continuer, confirmer modifie et etc. La loi l'arrivée de de 2016 hein qui qu'on skie. Renforcer justement le dialogue avec les supporters et qui visait notamment à lutter à l'époque c'était le terme contre le hooliganisme. Donc je dirais que c'est des dispositions que nous serons amenés semble-t-il à à débattre à nouveau entre nous, dans des textes à venir. Merci. Donc. Pour ce qui est de l'amendement. Je vais le soumettre aux voix avec un double avis défavorable. Donc il est pour. Tu es contre. Qui s'abstient. Il n'est pas adopté, je soumets aux voix l'article 13. Qui est pour l'article 13.

Merci, monsieur le Président Madame la Ministre, mes chers collègues. La Cour des comptes remettra son rapport définitif sur les jeux mi-2026 lorsqu'elle aura pu examiner les comptes définitifs. pardon oui cet article. Vise disposer dès 2025 noeuds rapport d'étape remis au Parlement qui permettra d'examiner une photographie des comptes afin de constater en particulier, le respect de l'équilibre du budget, compte tenu du temps nécessaire à la cour pour obtenir les données financières indispensables à la réalisation de ce bilan d'étape. Et du délai incompressible inhérents à la procédure contradictoire le présent amendement propose un accord avec la Cour de repousser repoussé au premier octobre 2025. La date limite de remise de ce rapport au Parlement.

Bien, donc un amendement présenté par le rapporteur et qu'un avis favorable du gouvernement, pas de demande d'explications de vote, qui est pour. Qui est contre.

Mesdames les ministres, mes chers collègues pour le bon déroulé des Jeux olympiques et par Aoun rue olympique. Les organisateurs comptent sur une mobilisation de 45.000 bénévoles, ils rempliront des missions essentielles d'accueil et d'orientation du public mais également d'assistance des athlètes et du personnel médical et encore des missions de logistique administrative. Cela pourrait constituer une très belle expérience intergénérationnelle pour des milliers de personnes comme seuls les expériences de bénévolat peuvent offrir. Mais afin que les jeux restent une fête pour eux aussi. Il nous paraît essentiel d'alerter les organisateurs sur la nécessité de leur aménager des conditions de mobilisation plus plus favorables que ceux qui n'est prévu. L'achat des bénévoles publié sur le site des Jeux prévoit notamment la possibilité de les mobiliser jusqu'à 48 heures hebdomadaires et 10h par jour en les défrayant seulement de frais de transport et d'un seul repas quotidien. Afin que toute la lumière soit faite sur leurs conditions de mobilisation. Nous proposons donc de donner mission à la Cour des comptes, d'en faire le bilan. Ah. A posteriori, faute d'avoir pu encadrer le temps de mobilisation dans ce texte. Si Madame de Marco et encore toutes mes excuses pour cet oubli monsieur le rapporteur. Oui, merci Monsieur le Président Madame la Ministre, mes chers collègues. Comme vous l'avez rappelé Madame de Marco. La question des bénévoles constitue effectivement un point de vigilance pour la réussite des Jeux. Il est donc essentiel de s'assurer que les bénévoles bénéficieront de toute l'attention qu'il mérite. C'est donc un avis favorable. Madame la Ministre. Un avis de sagesse. C'est en effet ce thème du bénévolat, point très important, mais il y aurait beaucoup d'autres points à couvrir, qui ne sont pas tous énumérer. Voilà, raison pour laquelle je rends cet avis de sagesse. Bien, donc je vais soumettre l'amendement voit avec un avis favorable de la commission un avis de sagesse du gouvernement qui est pour. Qui est contre. S'abstient-il être adopté. Donc je soumets aux voix l'article 14 A qui est pour. Qui est contre. Qui s'abstient. Il est adopté. Après l'article 14 à en première amendement le l'amendement numéro 15. Madame de La Gontrie. Merci, monsieur le Président. Madame la Ministre, mes chers collègues. Cet amendement. A vocation à permettre le pavoisement notamment concernant les JO, les 10 métropoles qui vont accueillir. Des événements et de permettre à cette occasion. Donc le pavoisement lors de grands événements sportifs internationaux pour rendre plus visible et permettre à l'ensemble des habitants de s'approprier ces ces manifestations, c'est évidemment à caractère exceptionnel mais il faut adapter le droit et donc ces événements. Concernés devraient être déterminée par décret. Et permettrait ainsi de rendre. Visibles et de. Pavoiser il y a pas de mot plus adapté les villes à l'occasion des Jeux olympiques. Merci monsieur le rapporteur. Merci, monsieur le Président Madame la Ministre, mes chers collègues. Cet amendement vise à rendre permanente les dérogations à la réglementation. Sur les publicités dans l'espace public à l'occasion des grandes manifestations sportives afin de permettre la mise en valeur des organisateurs et de leur sponsor. Il aurait en pour effet de porter atteinte de manière habituelle à la protection du Patrimoine alors que de nombreuses critiques ont déjà été émises par les sénateurs sur l'article 14 qui prévoit des dérogations exceptionnelles pour les Jeux olympiques et paralympiques. L'amendement numéro 36 de notre collègue de Marco appelle par exemple a supprimé l'article 14, afin de limiter les dérives commerciales. Concernant l'organisation de la Coupe du monde de rugby. J'indique que nous n'avons été saisis d'aucune demande de la part des organisateurs. On peut néanmoins remarquer que l'organisation de l'euro 2016 n'avait pas nécessité d'introduire des dérogations permanentes à la réglementation sur la publicité dans le code de l'environnement, donc c'est un avis défavorable. Madame la Ministre. du cadre de vie et j'ajoute, comme l'a fait le rapporteur, que ces éléments-là ne nous sont pas remontés comme des demandes de la part du mouvement sportif et des organisateurs de grands événements. Donc pour nous c'est retrait ou sinon Roger. Donc un double avis défavorable. Pas de demandes d'explications de vote, donc je le soumets, on voit qu'il est pour cet amendement. Qui est contre. Qui s'abstient. Qui n'est pas adopté. Après l'amendement 16 rectifié suspension. Merci, monsieur le Président Madame la Ministre chers collègues cet amendement tend à permettre aux collectivités dans lesquelles les festivals et autres événements festifs devront être reportées du fait de leur simultanéité avec les GOP et l'impossibilité d'assurer leur sécurité de pouvoir décider d'une anticipation ou de d'un report des dates de congés scolaires, au delà du cadre réglementaire autorisé de trois jours. Ainsi la tenue du festival d'Avignon par exemple va être. Et se tiendra à partir du 29 juin 2024. De nombreuses représentations de ce festival ont lieu dans des établissements scolaires. Il est absolument nécessaire de pouvoir avancer les vacances scolaires fixée pour le de 2024 au 6 juillet. Au delà des 3 jours réglementairement autorisée. Pour libérer les locaux de ces établissements pour les besoins de représentation et de répétitions des spectacles. Je ne comprends pas l'argument avancé par notre rapporteur lors de la commission il est nullement satisfait par la réglementation en vigueur, contrairement à ce qu'il a été affirmé l'article des 521 1 du code de l'éducation dispose les recteurs d'académie ont compétence pour procéder à des adaptations du calendrier scolaire national rendu nécessaire soit par la situation géographique particulière d'un établissement ou la nature des formations qu'il dispose dispense pardon, soit par des circonstances susceptibles de mettre en difficulté dans un établissement un département ou une académie le fonctionnement du service public de l'enseignement. L'article des 521 2 précise les dates des vacances des écoles maternelles et élémentaires peuvent être alignée sur celle des collèges du secteur auxquelles elles sont rattachées lorsque ce collège est implantée dans le territoire d'une académie appartenant à une zone de vacances différentes peuvent être modifiés, soit la durée soit seulement les dates d'une période de vacances inclus dans l'année scolaire. La date de la rentrée scolaire peut également être retardée. Ces modifications ne peuvent excéder 3 jours consécutifs. Il me semble donc que cet amendement est utile puisque puisqu'il prévoit des dispositions. Pour les festivals anticiper au reporter de 2024 qui ne rentre pas dans le cas prévu dans le code de l'éducation. En outre, la réglementation dont je viens de donner lecture ne concerne que les établissements du 1er degré. Donc je demande à la. Merci, merci chers collègue. Merci beaucoup, je crois qu'on a, on a compris le sens de votre amendement. Monsieur le rapporteur. Oui, merci Monsieur le Président Madame la Ministre, mes chers collègues. Je suis naturellement conscient de la difficulté. On en a encore parlé ce matin d'organiser certains festivals et. Il ne faut pas qu'on. Se faire affronter sport et culture. Et nous en sommes tous conscients, à ce niveau-là. Mais comme je l'ai dit c'est le. On peut déjà aujourd'hui. Adapter les congés scolaires par exemple, vous citez. Le festival d'Avignon pour le festival d'Union les congés scolaires

effectivement au au date nécessaire d'après eux mais. C'est le gouvernement peut dès dès aujourd'hui par non pas par la loi mais par voie réglementaire. Il peut adopter des aménagements qui lui semblent souhaitables pour. Répondre aux défis qui sont constitués par l'organisation des Jeux olympiques et paralympiques. C'est pourquoi je dis que cet amendement est satisfait. C'est donc une proposition de retrait ou un avis défavorable. Alors Madame la Ministre. Oui je dirais satisfait. Donc rejet dans la mesure où je là aussi je partage absolument votre approche pragmatique nous aurons probablement besoin de faire quelques ajustements sur ce registre. Mais précisément, nous sommes aujourd'hui en train de travailler avec Pap Ndiaye. Sur le décret qui va étendre la faculté d'adaptation des recteurs. C'est un décret, un décret pardon qui est en cours de, de préparation, qui sera publié dans les prochains mois et qui apportera la réponse aux besoins de vous identifier justement, on est là dans du ressort du réglementaire et non pas de la loi. Merci.

Qui s'abstient. Il n'est pas adopté. Maintenant l'amendement 41 Madame Marco. 227 millions d'euros dans un total du budget du COJOP qui s'est levé, alors un peu moins de 4 milliards d'euros. Il s'agit de l'enveloppe destinée je cite à assurer la neutralité totale des émissions de carbone liées à l'organisation des Jeux. Il y a conduire des politiques innovantes en matière d'excellence environnementale. Pourtant, le budget alloué à ce poste de dépense est inférieur à celui des relations internationales destinées à l'accueil des 200 délégations des comités nationaux, celui-ci était de 31,6 millions d'euros. On peut s'interroger sur cette répartition budgétaire si cela recouvre l'achat du billet d'avion pour les délégations, cela signifierait qu'il faudrait au moins que l'excellence environnementale soit égal à ce mental montant le compte n'y est pas. Afin d'augmenter les moyens nécessaires pour l'excellence environnementale. Nous proposons donc au gouvernement de réfléchir à l'instauration d'une taxe sur les produits dérivés vendus pendant les Jeux. Pour financer cette excellence environnementale. Monsieur le rapporteur. Et on a eu un. Débat en commission pour au moins 3 raisons, la première c'est que la billetterie des Jeux est ouverte et qui n'apparaît pas possible d'augmenter le prix des billets au travers d'une nouvelle taxe aujourd'hui. La 2ème c'est que le budget du COJOP, on le sait est fragile et il ne serait pas judicieux d'adopter une disposition qui aurait un impact sur ses recettes et la troisième c'est qu'une telle disposition aurait dû être adopté il y a un nous deux ans. Pour pouvoir être mises en oeuvre aujourd'hui. On peut néanmoins s'interroger sur le fond. Sur sa compatibilité avec les dispositions du contrat de ville hôte qui fixe le cadre du déroulement des Jeux dans les moindres détails. Il y a donc c'est un avis défavorable. Merci monsieur le rapporteur. Madame la Ministre. Avis également défavorable dans la mesure où on cherche vraiment à simplifier le droit fiscal à supprimer les taxes à faible rendement. On est évidemment très sensible à la manière d'utiliser ces produits dérivés, mais cette réponse de nature fiscale ne nous semble pas adaptée donc défavorable. a un double avis défavorable je soumets l'abondement voix qui est pour. Qui est contre. Qui s'abstient. Il n'est pas adopté. Nous passons aux amendements de l'article 14 Madame démarre. Merci. L'article 14 de la loi que nous examinons prévoit que les partenaires privés des Jeux puissent bénéficier des dérogations pour l'affichage de leur logo sur l'espace public. Il y a proximité des monuments historiques. 15 jours avant et 7 jours après le passage de la flamme. Dans le rapport, il est souligné que le parcours du relais de la flamme ne pourra concerner que des communes volontaires et qu'aucune dépense ne pourra leur être imposé le cours du relais de la flamme étant pris en charge par le comité d'organisation. Mais le passage de la flamme olympique va tout de même coûté au contribuable, 180.000 euros par jour versée par chaque conseil départemental des 60 départements traversés. Dans le même temps le secret des affaires ne nous permet pas de savoir ce qui sera à la charge des partenaires commerciaux. Nous nous opposons donc aux dérives commerciales dénaturant l'esprit des Jeux et surtout quand elle dénature aussi nos paysages et nos centre-ville par l'ajout de panneaux publicitaires. Nous proposons donc tout simplement la suppression de l'article 14. Merci Monsieur le Président Madame la Ministre, mes chers collègues, l'adoption de cet amendement de suppression reviendrait tout simplement à rendre impossible l'organisation du relais de la flamme et donc les Jeux olympiques et paralympiques elle mettrait également en faute la France vis-à-vis du CIO au regard des dispositions du contrat ville hôte. C'est donc un avis défavorable. Monsieur le président. L'avis défavorable pour les mêmes raisons. Et j'ajoute un cette conciliation que nous avons recherché et que le Conseil d'État a lui-même reconnu entre ses exigences tiré du contrat de ville hôte et la préservation du cadre de vie et de l'environnement. Bien double avis défavorable. Pas de demande d'explications de vote, je le soumets on voit qui est pour. C'est contre. Qui s'abstient n'est pas adopté ensuite trois amendements qui font l'objet d'une discussion commune. D'abord le 74 monsieur Dossus. Merci monsieur le président. On va revenir sur la publicité qui est. Autorisé à tort et à travers par. Cet événement, y compris à travers l'Arctique 14 de faire de ces dérogations et. Nous proposons d'encadrer un peu plus. Les dispositifs publicitaires puisque nous considérons que loin des valeurs de l'olympisme. Le texte nous propose ici de nous enfoncer encore plus dans la dérive mercantile et commercial de cet événement qui ne sert que de vitrine publicitaire à ses sponsors et donc nous avons une une opposition de principe à cet article puisque ma collègue vient de le le le défendent mais. Nous en proposons ici à un moment de repli qui qui qui qui vous permet d'encadrer un peu mieux cette publicité en. L'interdisant sur les supports panneau numérique. Sur le parcours de la flamme et sur le site du compte-à-rebours. En effet, la publicité lumineuse et surtout celle réalisée sur les panneaux numériques est une aberration écologique et le l'événement s'engage à à à être très responsables sur ce saut à ce niveau. On va rappeler que les calculs là, démontre que les panneaux numériques consomme autant d'énergie sur leur durée de vie que 4 ménages français en une année, donc ils sont extrêmement énergivores si on en croit la communication officielle les instances organisatrices des Jeux. Ceux-ci ont pour ambition d'être plus les plus écologiques de l'histoire avec cet amendement, je vous propose une mesure simple, efficace de bon sens pour tendre dans cette direction. Monsieur de. Je vous propose de présenter les deux suivants parce qu'ils sont tous les 3 en discussion commune. Donc le 60 15 et le 73. Oui le. Le 75, vise la même chose mais pour interdire la publicité sur les espaces verts puisque sont autorisés. Ça nous paraissait saugrenue. Donc c'est la même chose que mon précédent amendement mais sur les espaces verts C'est pour revenir sur l'article 5 de la loi JO de 2018 sur la publicité. Qui permettait donc comme l'article 14, un certain nombre de dérogations. Par exemple d'autoriser dans un rayon de 500 mètres autour de chaque site olympique. Ce qui au vu de la concentration des sites en Île-de-France représentent une surface considérablement. D'autoriser la publicité sur les immeubles classés les monuments historiques ou naturels et les sites patrimoniaux remarquables. C'est-à-dire que dans tous ces sites nous pourront voir s'afficher en grand des publicités pour des marques comme Coca Cola, l'un des pires pollueurs responsable. Cette entreprise est responsable de 10% des déchets plastiques dans le monde en émettant pour la production de ces bouteilles, 15 millions de tonnes de CO2 chaque année, soit l'empreinte carbone d'un pays comme le Cambodge qui pourra donc collé son nom sur les sites classés de notre pays puisque elle est partenaire du marketing mondial des jeux c'est incompatible avec l'ambition environnementale des JO. On nous dit on nous répète notamment dans la politique de l'hérite d'héritage des Jeux que si ceux-ci seront neutre en carbone et on apprend un emprunt thème positif sur le climat. Mais comment les citoyens et citoyennes pourrait y croire, ne serait-ce qu'une seule seconde en voyant fleurir dans leur ville des affiches immenses à la gloire des plus grands destructeurs de biodiversité. L'urgence n'est pas d'ouvrir plus d'espaces de publicité à ces entreprises, mais au contraire de les limiter, voire de les faire disparaître. C'est précisément le but de cet amendement. dessus. Monsieur le rapporteur. Sur ces trois amendements. Est une proposition de bon sens au regard de la crise énergétique que nous connaissons. Elle doit constituer une préoccupation des organisateurs qui sont déjà sensibilisés à l'impératif de sobriété énergétique, néanmoins il n'apparaît pas souhaitable d'inscrire cette interdiction dans la loi car elles pourraient contrevenir au contrat de ville hôte. Je souhaite quand même que ce sujet soit porté dans le cadre du dialogue institutionnel qui existent entre l'État, la ville de Paris et le COJOP, c'est donc un avis défavorable pour le 74. Le 60. 15 on peut là encore qu'être sensible au fait de préserver les espaces naturels des villes de de la publicité. Cependant, là encore il n'apparaît pas judicieux de prévoir cette interdiction dans la loi. Il faut savoir qu'au niveau de chaque commune maire conservera la poupée possibilité d'autoriser ou non les affichages dans le cadre de son pouvoir de police générale, c'est donc également un avis défavorable. Et enfin l'amendement 73. L'adoption de cet amendement remettrait en cause gravement le respect du contrat de ville hôte et reviendrait sur les engagements pris par notre pays pour accueillir les Jeux, c'est donc également un avis défavorable. Merci, madame la Ministre, sur ces trois amendements. Même avis défavorable je préciserai juste hein par rapport à ce que vient d'exposer le le rapporteur, que le dispositif qui vous est proposé, il exclut déjà du chant des dérogations, les publicités numériques. Ça c'est un 1er point, s'agissant des affiches qui sont éclairée par projection ou par transparence. Une déclaration préalable et nécessaire auprès de l'autorité de police compétentes et cette autorité de police peut tout à fait s'opposer à l'installation ou bien la subordonnée au respect de conditions qui seraient par exemple destinés à préserver l'insertion architecturale paysagère et donc il y a déjà ses garde- fous qui sont tout à fait prévues par le dispositif et pour le reste nous sommes tenus par les engagements du contrat de ville Bien, donc un double avis défavorable sur les trois amendements que je vais donc soumettre aux voix. Donc l'amendement 73. 74 pardon le 1er 74 qui est pour. Qui est contre. Qui s'abstient. Il n'est pas adopté le 75 même botte. Vote le 73 même botte. Même vote, donc ils ne sont pas adoptés je vais soumettre aux voix l'article 14 qui est pour l'article 14. Qui est contre. Qui s'abstient. Il est adopté. Après l'article 14 l'amendement 37 madame Marco. Comme vous le savez, la saison estivale est aussi la saison des feux de forêt comme ceux qui ont ravagé celle de La Teste du bus et de Landiras en Gironde l'été dernier à Bordeaux, nous serons ravis d'accueillir des spectateurs des épreuves olympiques de football mais il n'aime pas d'être vigilant quant à la prévention des risques liés au tourisme de masse pour la biodiversité. Et aux écosystèmes fragiles que sont les forêts en été. Il en avant. De même dans d'autres territoires qui accueilleront des épreuves et pour d'autres écosystèmes. Je lis dans le rapport de la Cour des comptes déjà cités que 17 6 millions d'euros du COJO sont affectés à la communication 50 millions à l'impact et à l'héritage de 102 millions à la marque aux événements et aux cérémonies. C'est pourquoi, afin de permettre la bonne information des spectateurs des Jeux. Je propose qu'une fraction de ces Budgets soient affectés à l'information de spectateurs tous les risques de l'activité touristique annexe pour la biodiversité, environnement. Merci, monsieur le Président Madame la Ministre, mes chers collègues. Cet amendement des. Rappelle l'importance des messages au public afin de protéger l'environnement. Si l'objectif est louable et partagé, il n'apparaît pas judicieux d'inscrire ce principe d'information dans la loi, compte tenu du fait que l'organisation des Jeux a été défini précisément dans le contrat de ville hôte. C'est donc un avis défavorable. Même avis monsieur le président. Et j'ajouterai juste que le comité d'organisation a lui-même pris cet engagement d'en effet promouvoir ses messages de prévention ces écogestes auprès de l'ensemble des spectateurs et nous y veillerons de manière rigoureuse.

Donc je vais soumettre aux voix l'amendement l'amendement 37 qui est pour. Qui est contre. Qui s'abstient. N'est pas adopté. Donc après l'article 14 à nouveau l'amendement 38 Madame de Marco. Ça, ça nécessitait pas un scrutin public pour mais bon. J'aimerais bien savoir pourquoi. À priori on vote contre l'amendement précédente par exemple. Mais écoutez, j'ai pas d'explication de vote comme je l'évoquais précédemment, l'excellence environnementale, la politique d'héritage font figure d'angle mort dans la préparation de ces Jeux. Même le le rapport de la Cour des comptes est relativement lacunaires leurs propos. Nous disposons actuellement de peu d'éléments pour pu juger de l'avancée des engagements du comité organisateur, en matière de préservation de la biodiversité et d'émissions de gaz à effet de serre. Le droit français prévoit des mesures de compensation en cas en cas d'atteinte à la biodiversité. Et c'est également la politique environnementale semble-t-il retenu par le comité organisateur. Nous aurions préféré des mesures de prévention. En lieu et place de mesures de compensation il nous aurions souhaité un suivi plus détaillée, se disant peut-être atteinte constatée ou anticipée. Afin de pouvoir toutefois évaluer l'efficacité des mesures de compensation. Annoncée. Nous proposons donc par cet amendement de produire une publication annuelle retraçant ces mesures. Merci cher collègue là monsieur le rapporteur. Oui, merci monsieur le président, madame la ministre, mes chers collègues. Cet amendement vise donc à imposer aux organisateurs des Jeux la publication annuelle des mesures de compensation. Outre le fait qu'une telle obligation pourrait contrevenir au contrat de ville hôte, il convient d'indiquer que l'adoption de cette mesure aurait dû être fait dans une prison précédente loi consacrée aux Jeux olympiques et paralympiques afin de prévoir justement le temps nécessaire à la mise en oeuvre d'un tel dispositif. C'est donc un avis défavorable. Madame la Ministre. Seront les plus écologiques de l'histoire avec un engagement inédit qui a été pris par le comité d'organisation de diviser par 2 les émissions de gaz à effet de serre et d'avoir même une neutralité carbone grâce à des investissements de plusieurs millions d'euros dans des projets de soutien à la biodiversité. Sur la traçabilité de ses engagements. Un rapport dédié et publié sur le site du comité d'organisation Paris 2024, un rapport qui est intitulé durabilité héritage une première édition de ce rapport a été publié en juillet 2021, d'autres éditions suivront et trace de manière détaillée. Le détail des mesures d'évitement de réduction d'impact ont été mises en place ainsi que les estimations d'impact carbone et le programme de compensation qui est déjà déployé un 2ème rapport sera publié au printemps 24 et un 3e, juste après les Jeux. C'est vraiment une dimension sur laquelle nous sommes très engagés, et rendront des comptes. Bien, merci madame la ministre monsieur Ouzoulias. Merci monsieur le président, ma Madame la Ministre vous vous venez de faire une déclaration forte, les jeux olympiques seront les les plus écologiques de de l'histoire des Olympiades. Moi j'aimerais revenir sur le problème des réseaux de transport alternatifs. Il y avait quatre lignes de transport de métro qui a qui qui était prévu dans le cadre de la candidature. Ils ne seront pas réalisées. Et vous allez mettre en place 1700 bus tous les jours. Est-ce que je dois comprendre de votre déclaration aujourd'hui que ce sont tous des bus électriques et dans ces cas-là vous m'expliquez ou vous allez trouver les bus et ensuite les chauffeurs. Merci monsieur le président. vous avez raison, Monsieur le Sénateur, de rappeler que tous les projets d'aménagement qui avait été. En son temps en leur temps annoncé dans la phase de candidature n'ont pas pu être réalisés pour des raisons de soutenabilité budgétaire parfois aussi de calendrier de ces travaux. En revanche, je pense à l'axe de la ligne 14 qui va être absolument essentiel au sud, Orly au nord, la gare de Saint-Denis Pleyel les travaux les travaux également qui sont effectués autour d'Eole. Donc notre réseau de transports en commun restera le point absolument névralgique de toute la desserte pour nos jeux olympiques et paralympiques. Nous avons également prévu oui. L'utilisation d'un certain nombre de véhicules hybrides. Ça fait d'ailleurs partie des engagements que nous avons dans le cadre des partenariats qu'on appelle Top avec Toyota qui est l'un des sponsors principaux du CIO, vous l'avez en tête et je voudrais aussi bien entendu souligner compte tenu de l'engagement du gouvernement sur la question du vélo l'effort très important fait sur l'ensemble du réseau de voies cyclables le déploiement de stationnement de vélo et tout le travail que nous menons pour que l'ensemble du maillage nous permettent de bien desservir l'ensemble des sites de compétition dans les meilleures conditions de préservation de l'environnement. Merci. Nous allons maintenant passer au vote sur le l'amendement. Numéro 38 avec un double avis défavorable qui est pour. C'est contre. Qui s'abstient n'est pas adopté nous passons l'article 15. Avec l'abondement 54 madame Gréaume. Merci monsieur le président, madame la ministre. L'article 15 prévoit que les fonctionnaires occupant un emploi supérieur les conduisant à participer directement à l'organisation des Jeux de Paris 2024. Peuvent rester en fonction au delà des 2 ans prévus par la loi. Jusqu'au 31 décembre 2024. Bien entendu, avec l'accord des personnes. La limite d'âge des fonctionnaires ou coupants un emploi supérieur est fixé à 67 ans. Le gouvernement veut donc au nom de l'intérêt du service maintenir en activité des fonctionnaires au-delà de 69 ans. Souhaite le gouvernement reconnaît que les politiques de non remplacement des départs en retraite de la fonction publique entraîner un affaiblissement des capacités de pilotage public et une perte de savoir-faire. Souhaite le gouvernement doit assumer que les jeunes ne serait pas capable d'organiser les Jeux olympiques et paralympiques. Et dans ce cas, ils devront en faire la démonstration. En attendant cette mesure dérogatoire même limitée dans le temps et pour les personnels concernés n'en demeure pas moins une dérogation à l'âge maximal de travail et in fine et une remise en cause du droit à la retraite, alors même que le gouvernement a présenté hier son projet de loi de réforme des retraites des retraites qui allonge à 64 ans l'âge légal de départ en retraite et allonge le nombre d'annuités à 43 ans. Nous refusons totalement cette mesure pour ces raisons, nous demandons la suppression de cet article, merci. Merci cher collègue. Madame la rapporteure. Oui, monsieur le président, madame la ministre, mes chers collègues. Alors ce sera pour cet amendement un avis défavorable cet article 15, vise à prolonger effectivement. Les

à l'organisation des Jeux olympiques et para-olympiques. Il est vraiment dans la cible du projet de loi, c'est pour ça que nous. Pensons que dans l'intérêt de cette organisation dans le l'intérêt du bon déroulement des Jeux olympiques, il convient en toute logique de maintenir le préfet jusqu'au terme de l'organisation de ces Jeux olympiques, donc c'est un avis défavorable. Madame la Ministre. Peut-être mon retour d'expérience sur la vaste Titudes de ce que nous avons réalisé en terme d'organisation autour de ces Jeux olympiques et paralympiques et la courbe d'apprentissage que tout ça suscite la somme de détails de boulons à serrer sur l'ensemble des dimensions. Le transport, la sécurité, toutes les mesures héritage la préparation de l'écosystème autour de nos athlètes, les différentes dimensions d'articulation avec les territoires pour faire en sorte que que ces je puisse bénéficier à tous les Français, c'est d'une immense complexité d'une immense difficulté nous avons vraiment besoin dans cette aventure humaine de garder. Les personnes les plus expertes les plus engagés et de les laisser aller au bout de cet exercice pour faire réussir la France. Monsieur Ouzoulias. Monsieur le Président Madame la Ministre j'ai j'ai bien entendu ce que vous nous avez dit madame la la rapporteure donc. Si il s'agit que d'un seul fonctionnaire il faut rectifier votre votre texte de loi qui dit, pour tous les fonctionnaires et enlever le pluriel pour le fonctionnaire et ça sera beaucoup plus clair pour tout le monde. Merci monsieur le président. Madame la Ministre. Qui sont nécessaires autour de de de cela, c'est vraiment la personnalité la plus emblématique, Michel Cadot prenant évidemment. Une importance particulière dans le pilotage de cette action de préparation des Jeux. Bien merci. Nous allons donc passer aux voit sur cet amendement avec un double avis défavorable qui est pour cet amendement le 54. Qui est contre. Qui s'abstient. Il n'est pas adopté. L'amendement 55. Monsieur Ouzoulias. Merci, monsieur le Président Madame la Ministre. Comme le préfet cadeau va être extrêmement mobilisés sur les jeux nous nous proposons de prendre des vacances plutôt. le souhaitez, de prolonger la dérogation jusqu'au 21 décembre. Nous, on propose de la prolonger jusqu'à la fin du mois de septembre comme ça, ça permettra aux préfets cadeau de se reposer. Je pense que il aura tout à fait mérité ce ce congé supplémentaire. Merci monsieur le président.

après l'organisation des Jeux olympiques. Il faut faire derrière l'évaluation donc non. 31 décembre et on n'est contre et donc c'est un avis défavorable. Madame la Ministre. Défavorable pour les mêmes raisons. Et j'ajouterai que le préfet cadeau est particulièrement attentifs à cette dimension d'évaluation il a mis en place une méthodologie autour de 13. D'évaluation très précis qui nous permettront de mesurer les impacts économiques, sociaux, ainsi que l'effet des mesures d'héritage pour essayer de faire de notre pays une nation plus sportive. Monsieur Kader. Oui, monsieur le Président Madame la Ministre. Nous ne voterons pas d'amendements apportés par nos collègues communistes. Voteront contre, parce que ce cadeau est connu de beaucoup d'entre nous. C'est un très grand serviteur de l'État. C'est l'objet, c'est l'efficacité de. Madame Assassi je vous remercie de me laisser parler. La la la question qui est posée c'est, quelle est la meilleure personne pour assurer les fonctions qui sont déterminés par. Les priorités évoquées par Madame la Ministre. Ce credo a suivi ce dossier depuis le début. Grand serviteur de l'État. Et pour ce qui me concerne une moi qui ai travaillé avec le préfet Lambert sur l'organisation de l'euro 2016 qui était aussi. Limite au niveau de l'âge, je considère, je considère que. Lui permettre d'aller jusqu'au bout de sa mission est un plus pour l'organisation de ces Jeux olympiques, je voulais quand même le souligner parce que il est bon de temps en temps de dire du bien des grands préfet qui aujourd'hui comporte. Et valorise l'image de notre pays. Madame Groux. Non c'est bon. Bien, donc je vais soumettre aux voix cet amendement avec un double avis défavorable qui est pour. Qui est contre. Qui s'abstient. N'est pas adopté. Un amendement présenté par Monsieur Patriat. Merci. Monsieur le président. Merci. Mes chers collègues. Cet amendement a pour but de permettre aux dirigeants d'établissements publics en fonction à la date d'attribution des Jeux olympiques et paralympiques et participant directement à leur organisation de pouvoir continuer à exercer cette fonction jusqu'à la fin de l'année 2024. Nonobstant toutes disciplines Cette mesure générale concernent notamment la présidence de l'établissement public du château et du musée et du domaine national de Versailles. Qui comme vous le savez, accueillera les épreuves d'équitation et de pentathlon moderne l'actuelle présidente de l'établissement public a été nommé le 31 août 2011, elle a été reconduite 2 fois son dernier mandat s'est achevé en octobre 2022 la conduisant à exercer son propre intérim afin d'assurer la continuité de la gestion de l'établissement public et notamment son implication dans la préparation des Jeux olympiques. La poursuite de cet objectif conduit à déroger à 2 paramètres à savoir le nombre de mandats et la limite d'âge j'entends bien la solution réglementaire n'étant pas envisageable. La piste législative et c'est la privilégier. C'est la raison pour laquelle je vous invite à voter cet amendement, je vous remercie. Merci madame la rapporteure. vise directement la situation de Madame Pégard qui est à la tête. De l'établissement public du château de Versailles. On voit bien les difficultés qu'il y a aujourd'hui. C'est que passer par la voie législative est une issue sur laquelle nous émettrons un avis de sagesse. Monsieur le président. Et messieurs les sénateurs. Et madame. La rapporteure je je je vais m'appuyer sur ce que j'ai dit précédemment. En soulignant d'abord que les épreuves mentionné par François Patriat sont importantes on peut y rajouter aussi les épreuves de para-équitation ce site et parmi les sites peut-être le site le plus iconiques de l'organisation de ces Jeux olympiques et paralympiques sur lesquels l'attention du monde et ce que nous avons essayé de faire, c'est-à-dire d'avoir à la fois cette logique de compacité dans les équipements et en même temps de marier le sport au coeur de notre Patrimoine culturel est absolument. Centrale Centrale 3ème élément que je voudrais mettre en avant, c'est que à voir aux commandes de l'établissement, une personne qui en connaît les moindres recoins qui en connaît les difficultés d'aménagement, la nécessité de concilier l'agenda sportif avec les éléments de Patrimoine d'avoir une organisation logistique et des services qui soit à la hauteur de ce rendez-vous qui sera complexe à opérer. C'est un atout dans notre préparation. Ce que je voulais simplement également ajouter c'est que nous avons déjà dans les propositions, la proposition qui vous est présentée, elle n'a pas un caractère exceptionnel au sens où des établissements culturels déjà comme l'Institut du monde arabe comme notre dame n'impose pas de limite d'âge de limite en nombre de mandats et que il y a déjà eu des extensions. Je pense à ce qui s'est passé également à la Philharmonie avec Laurent Bayle sur l'extension à 70 ans, mais surtout le dernier point que je voulais mentionner c'est Madame Catherine Pégard évidemment ne fera pas que les Jeux olympiques et paralympiques dans la poursuite de ce mandat, si vous donnez ce cette autorisation. Mais elle le rôle qu'elle va jouer va être pour nous extrêmement important et est-ce un atout pour nous d'avoir une personne qui connaît tout cela qui a été à la barre de cette organisation de la négociation contractuelle de la mise en place des besoins des Jeux olympiques. La réponse est évidemment un grand oui en lettres capitales. Merci. J'ai plusieurs demandes d'intervention monsieur noirs. Merci monsieur le président. C'est pas une explication de vote serait plutôt une explication d'amendements de. Les motivations de cet amendement parce que je je je comprends pas bien, il y a des choses que je ne comprends pas bien dans les les arguments qui ont été déployés tout à l'heure par Monsieur Patriat. Est-ce que je, j'ai évidemment aucun doute sur les compétences sur la la plus-Value que peu. Provoqué le maintien des personnes. Que vous avez cité au poste qu'ils exercent. Depuis 2011, vous avez dit mais, mais 2 interrogations sont premièrement à leur date de nomination et ce qu'il y avait une méconnaissance de l'âge des personnes. 2ème question, est-ce qu'il y avait une méconnaissance de la date des Jeux olympiques. Est-ce que comme à Tokyo les les Jeux olympiques ont été repoussées ou est-ce que finalement ils vont se dérouler en 2024 et qu'il était prévu que ça se déroule en 2024 dans ce cas je je je trouve pas, il y a une sorte de contradiction dans les arguments que vous avez déployé c'est le l'objet tu nous on intervention je voudrais Merci monsieur Ouzoulias. C'est le président, madame la ministre. Encore une fois un cavalier c'est plus un, un projet de loi c'est un concours équestre. Alors je sais que les épreuves hippiques vont se débrouiller à à Versailles, mais quand même quand même. Là il s'agit de la présidente d'un établissement public dont la limite d'âge a été dépassé depuis 2021 le ministère de la culture n'a pas réussi en 2 ans à former quelqu'un qui puisse lui succéder pour prendre en charge la totalité des des épreuves. Il y a un souci. Je pense que les candidats manquent pas moi je peux vous en trouvez vraiment. À l'appel sur sur le fond, il est quand même tout à fait anormal que ces limites d'âge elles concernent généralement seulement le domaine de la culture toujours le domaine de la culture comme si le domaine de la culture pouvait échapper par une forme de de miracle à toutes les lois qui qui impose en francs en France de de façon extrêmement judicieuse. Les les limites d'âge alors ça a été le cas pour Notre-Dame avec le général Georgelin s'est de nouveau le cas ici. Peut-être que le ministère de la culture et c'est c'est quand même ce qu'a voulu Malraux soit un vrai ministère qui fonctionne comme les autres et qui évite systématiquement de travailler. Avec des dérogations législatif. Merci monsieur le président. Madame Robert. Oui, merci Monsieur le Président Madame la Ministre alors moi je vais un peu répété ce qu'ont dit mes collègues mais d'abord je voudrais que on on s'exprime devant c'est un moment qui est quand même un vrai cavalier législatif là quand même il faut se le dire et même la rapporteure là exprimé d'autre part, que penser de cet amendement si ce n'est, qui vient régler une situation. Que le président que le gouvernement a essayé de régler, via un décret. Que le Conseil d'État a retoqué à l'unanimité. Il faut quand même là aussi qu'on se le dise. Et comment le qualifier cet amendement moi je pourrais qualifier du fait du prince. Parce qu'à un moment la jurisprudence Georges là où notre dame de Paris. On va en avoir de nouveau, donc je crois que sous couvert si c'est. Sous couvert des Jeux olympiques. Il s'agit de régler une situation que je trouve ubuesque qui veut que. Cette présidente d'établissement public est en intérim depuis 18 mois. Alors c'est vrai que notre collègue Pierre Ouzoulias. Cela dit et qu'elle aurait pu éviter effectivement remplacé dans les règles de l'art. À ce moment-là. Alors. Je suis un peu triste de vous dire ça mais je trouve que le procédé n'est pas correct parce que c'est renvoyer une responsabilité du gouvernement au Parlement et nous prenons aujourd'hui c'est très seront politique qui n'est pas la nôtre. Donc, non seulement je ne je ne trouve pas ça correct je ne trouve pas ça exemplaire comme l'a dit le président Macron c'est très public qualifiée d'exemplaire. Je ne trouve pas ça je si j'étais triste et Pierre Ouzoulias. Cela dit, c'est qu'un moment on observe la phlébite ment du ministère de la culture qui auraient dû qui aurait pu remplacer Madame Pégard et vraiment dans mes propos, je n'ai pas envie ni de parler de la présidente, ni de faire son bilan. Ce n'est pas le sujet, ce n'est pas le lieu vous voyez bien que c'est la question du principe de procès de ce procédé qui nous met tous dans la difficulté et qui nous renvoie à une responsabilité qui n'est pas la nôtre.

Il est vrai que les épreuves qui vont se passe à Versailles sont importantes mais cette situation elle est connue depuis des années et et il est incompréhensible que il y a pas eu la préparation pour former quelqu'un pour prendre la suite. La date des Jeux olympiques est connu depuis des années la situation de cette personne est connu depuis des années, rien n'a été fait. Moi je suis je partage tout à fait les propos de de Sylvie, Sylvie Robert. C'est vrai que c'est plus un cavalier. Ça, c'est le fait du prince, ou de la princesse, mais voilà la situation. Et puis lorsqu'on veut. Moraliser la vie publique dans les discours, lorsqu'on veut vouloir replacer l'intérêt général en prix priorité et vouloir promouvoir la République exemplaire. On propose pas des amendements comme celui-là donc à titre personnel, je voterai contre. Monsieur le président. Je serais presque tenté d'être séduit par ce cavalier et et d'ailleurs vous êtes personnellement concerné parce que je serais tenté de le sous-amender si mon sous-amendement n'était pas. Anticonstitutionnel peut être alors ça serait peut-être un sous-amendement d'appel parce que je pense que le Sénat participe aussi activement à l'organisation scènes des Jeux olympiques et que les sénateurs, notamment celui d'Île-de-France. Donc vous faites partie, ce sont des éléments essentiels dans cette organisation et peut être que si le gouvernement proposé au Sénat un report des élections sénatoriales qui concerne au moins au moins. Peut-être que nous aurions un intérêt à étudier ce sous-amendement parce que dans ces conditions je me laisserai peut-être séduire alors. Je veux bien que toute la France ayant étant Ça pourrait s'étendre à l'ensemble du territoire national, mais j'attire votre attention que pour l'île de France. Je pense que nous prenons notre part nous parlementaires à l'organisation de ces Jeux et si on veut, qui se déroule comme notre rôle est essentiel. Il faudrait que le gouvernement envisage le report des élections sénatoriales. Monsieur Folliot. Merci monsieur le président. C'est pas la première fois que nous nous trouvons face à une telle situation ou un amendement. Vient sur un texte avec le lien à la limite. Toute de ce qu'. On peut appeler un cavalier législatif pour reprendre les propos de nos, de nos collègues pour autant. Moi j'ai écouté vos propos Madame la Ministre et ceci m'ont convaincu par rapport à un élément qui me paraît être un élément essentiel et fondamental, c'est le fait que nous sommes. moins de 2 ans de ces jeux olympiques et que par rapport à cela. Devons. Mettre en avant un seul point, il y a un seul élément, c'est celui de l'efficacité est aujourd'hui. À l'occurrence par rapport à. La présidente de l'établissement public de de de Versailles, elle est en charge de l'organisation d'un certain nombre de d'épreuves On peut dire qu'effectivement les choses auraient pu être traitées avant et notamment au regard d'un certain nombre d'un jeu d'éléments qui ont été dit par un certain nombre de collègues de manière tout à fait juste. Au regard du ministère de la culture. Mais la situation aujourd'hui, elle est celle-là. Et la question de, c'est de savoir comment on en sort et donc une l'opportunité qui nous est donnée dans le cadre de de cet amendement, c'est de trouver une issue à cette situation d'autant plus que la personne concernée je pense fait l'unanimité, par rapport à professionnalisme qui est le sien à la qualité du travail qui a été le sien au au sein de cet établissement public et Si Versailles. Va jouer un rôle important en termes d'accueil donc d'un certain nombre d'épreuves va contribuer aussi comme nombre d'autres établissements culturels dans notre pays au rayonnement de notre pays et à l'attractivité de ces Jeux olympiques c'est pour cela que je crois que nous devons essayer d'être raisonnable et la raison en l'occurrence pour moi c'est de voter cet amendement. Merci, monsieur le Président Madame la Ministre chers collègues je je pense que la République exemplaire est un slogan qui doit nous rassembler et je dois vous dire en écoutant les arguments que si le succès des jeux Olympiques tient au maintien dans son poste de la présidente de l'Établissement public du château de Versailles. Je suis préoccupé et je propose qu'on ajoute à l'amendement de notre collègue Patriat un dispositif de soutien et d'accompagnement pour veiller qu'elle ne puisse pas avoir aucun souci d'ici la tenue des Jeux olympiques, un accompagnement, une surveillance de la santé parce que vous le savez. Il n'y a pas de gens irremplaçables. Il y a des postes et je veux en profiter pour dire mon soutien aux préfets cadeaux et ma volonté effectivement traduite dans le vote qu'il puisse continuer sa fonction il y a des postes dont je ne pense pas qu'il soit absolument indispensable à la réussite des Jeux olympiques et s'ils le sont, c'est tout de même très dommage de se le dire au moment où le délai de grâce est passé voilà 18 mois que ce sujet est connu voilà 18 mois qu'il y a un intérim qui dure je ne comprends pas mais très franchement je ne comprends pas que le gouvernement n'anticipe pas une situation comme celle-là donc face à cette incompréhension et à l'exigence d'exemplarité pour ma part, je voterai contre cet amendement.

On évoque aussi beaucoup aujourd'hui les difficultés des seniors dans le travail, hé bien moi je crois qu'il faut encourager les seniors à pouvoir travailler plus donc je soutiendrai dès demain. Cet amendement. Quel dommage parce que tout se passait bien, sur ce texte. Jusqu'à présent. Et c'est un peu dommage que nous soyons dans une situation là. De complexification pour. Un amendement qui n'a pas un lien. Il faut bien le reconnaître très fort avec les, les Jeux olympiques. Moi je voudrais. Juste attirer l'attention de l'auteur de l'amendement en disant que la sagesse. Et peut-être de le retirer à ce stade. Si j'entends bien les positions des uns et des autres. Il est probable qu'il ne passe pas. Et à ce moment-là ça rendra. La poursuite du dialogue et de la discussion qui me semble nécessaire. Sur ce point, plus complexe. C'est pour ça. Monsieur le Président Patriat que il me semble qu'une solution au point où nous sommes arrivés serait peut être de retirer l'amendement. Nous pourrons nous saisir au niveau de la commission culture puisqu'après tout, on nous demande aux parlementaires de se saisir de cette question de la nomination. La présidence de Versailles, à ce moment-là peut être auditionnés. La la personne en question et dans le cadre du processus législatif puisqu'il y a passage à leur assemblée nationale qui aura probablement en CMP la question pourra se reposer mais dans des termes plus serein et mieux penser que la façon dont cet amendement est arrivé. Bien. J'ai plus de demandes d'intervention. Monsieur Patriat, vous voulez réagir à cette demande ou enfin nous dire si vous maintenez l'amendement. Mais j'ai j'ai bien compris que cet amendement pouvaient maître-certains dans le Bas-Rhin. Je ne ferais pas ce que font beaucoup de nos collègues de polémiquer parfois inutilement sur beaucoup de sujets, je renvoie de part et d'autre le passer sur d'autres cas de ce genre qui ont été votées sous l'influence de telle ou telle dans d'autres législature, je leur ferai pas être un jour là je leur dirai pas j'ai essayé de dire que la simplement. Versailles, c'est quand même un objet hors du commun qui se dirige pas comme ça du jour au lendemain. La préparation a été commencé par une personne je demande simplement que la personne qui a commencé. Puisse le poursuivre s'agit pas de répondre à telle ou telle puis je dirais. Monsieur le Président la font que il suffit je j'ai pas besoin de retirer le il suffit qu'ils votent pour l'amendement avec ses amis pour que j'ai pas le retirer. Voilà, merci. Donc il est maintenu monsieur de. Merci monsieur le président, cher collègue. Une une simple explication de vote. J'ai le lait. L'occasion en discussion générale. D'exprimer l'hostilité du groupe Union centriste à la méthode. de rappeler que l'état de droit. Le fondement de l'État de droit. Le fondement de la démocratie, c'est le respect de la règle même quand elle n'arrange pas. Et la changer par différents moyens. Finalement. Objet d'une réprobation du Conseil d'État ou par un amendement cavalier comme ça a été dit sur plusieurs bon ne nous sommes pas à la, à la hauteur du travail que nous avons amené parce que finalement nous délibérons en tant que législateur sur l'opportunité de maintenir ou pas une personne en fonction. Au mépris des règles qui prévalait c'est ça ce que nous sommes en train de faire, de manière générale et absolue. C'est donc le groupe Union centriste, a exprimé farouchement son hostilité à la méthode. Maintenant. Nous avons en tête aussi qu'il s'agit d'une compétence. Gouvernementale. Et qui ne nous appartient pas de porter la charge. D'adopter ou non cet amendement et donc la majorité du groupe. A comme position il y a quelques votes hostiles quelques vote d'adhésion à l'amendement mais la majorité du vote du du groupe A. Comme position de renvoyer le gouvernement et et ceux qui le soutiennent. Par le, le, le dépôt de cet amendement ou une adhésion à cet amendement à ses responsabilités, ce n'est pas notre travail de législateur, c'est celui du gouvernement et donc nous renvoyons à l'auteur de l'amendement et à ceux qui souhaitent se positionner en tant qu'acteurs gouvernementaux et pas en tant que législateur de prendre la décision, en lieu et place du gouvernement.

la dernière datait de 2018, qui était antérieur au 2ème renouvellement de Catherine Pégard. Donc je voulais juste rectifier ces ces 2 éléments là qui ne change pas les positions qui ont été exprimées et simplement pour qu'on peut conclure sur ce point là ce que je peux vous dire d'un strict point de vue des besoins opérationnels des Jeux, nous serons plus forts avec Catherine Pégard demain. Président Patriat. Sur le terrain. L'amendement est retiré nous allons voter. Sur l'article 15. Qui est pour l'article 15. Qui est contre. Qui s'abstient. Il est adopté. Article 16. L'amendement 77 monsieur Dossus. Merci monsieur

l'organisme d'aménagement du territoire de la région. Île-de-France, la question de cette fin de vie est centrale, car les J. O. P de 2024 ont affiché l'ambition extrêmement élevé. Vous l'avez rappelé plusieurs fois lors de l'examen de ce texte en matière de durabilité et d'héritage ambition qui devra contrit continuer à produire des effets bien après les Jeux. Toutes les parties prenantes aux JO, dont Solideo fait partie en 1er chef ont signé le plan Héritage et durabilité, qui comporte des engagements extrêmement forts neutralité carbone des Jeux contribution positive au climat améliorer l'offre sportive dans le Nord-Est parisien structurer les filières et métiers du sport transition environnementale des événements sportifs, développement de l'offre sportive territoriale voilà des objectifs importants de long terme et qui engage fortement les signataires au 1er rang desquels on retrouve Solideo ainsi avant la fusion avec GPA, il nous semble légitime de dresser un point d'étape, un bilan de ses engagements afin de voir ce qui a été fait et ce qui reste encore à accomplir. Nous souhaitons ainsi que, au plus tard le 31 décembre 2025 Solideo rendre un rapport complet sur son action en matière d'aménagement et d'infrastructures ne souhaitons aussi qu'un point d'étape détaillées en matière de. De résultats sur les engagements écologiques fournis avec soit fourni avec ce ce ce document. Nous voulons également connaître la situation financière précise de cet organisme ainsi que les que des autres parties prenantes dans les actions qu'il mène souhaitant également savoir la manière dont Grand Paris Aménagement reprendra le flambeau. De cette mission héritage enfin, nous souhaitons que ces informations soient rendus publics car nous parlons ici 2 projets d'importance nationale qui influeront sur la politique sportive française pour les années à venir. Je vous remercie. Merci madame la rapporteure. et où c'est savoir seront transmis à Grand Paris Aménagement et nous ça pense à mener des garanties supplémentaires, donc nous émettons un avis favorable. Madame la Ministre. de. De sagesse dans la mesure où je comprends absolument et partage cette envie ce besoin de transparence financière. En revanche, ce que je voulais bien préciser, c'est que de 2026 à 2028 la Solideo va s'appuyer sur GPA mais conserver son propre budget, les établissements ne sont pas fusionner et la Solideo va vraiment garder ses comptes, son portefeuille d'activités, son budget, donc ça n'est pas une date absolument charnière au regard de cette trajectoire Pas absolument indispensable, me semble-t-il. Merci donc un avis favorable de la commission un avis de sagesse du gouvernement Monsieur de ballonné. Merci monsieur le président, chers collègues. Pendant l'intervention de notre collègue dessus. Et mon intervention est un rappel au règlement et ne demande d'excuses. Pendant l'intervention de notre collègue le président Patriat a fait ce signe suivant. J'espère que c'est enregistré. Avec une lecture sur les lèvres, on va te buter. J'ai demandé une précision et le président m'a a bien voulu m'indiquer à haute voix. Dans six mois tu ne seras plus rien pour confirmer son geste. Alors, je remercie le président Patriat qui veut me buter. Je note que nous n'avons pas buter son amendement pour reprendre cet élégant Champ lexical. Mais que nous l'avons peut être rendue possible et donc. À défaut d'avoir l'expression d'une gratitude du président Patriat je lui demande au moins des excuses.

tout ça. Cet incident est clos. Pour le moment vous continuerez vos explications hors de la séance. nous allons continuer donc voté sur l'amendement. 77 rectifié de monsieur Dossus avec un avis favorable de la commission à la ville sagesse du gouvernement qui est pour.

Qui est contre qui s'abstient il est adopté les articles 17 et 18 ont été précédemment examiner donc nous passons à l'amendement 76, après l'article 18 monsieur Bena. Merci monsieur le président. C'est vrai, je ne sais pas qui a dit tout à l'heure que tout s'était très bien passé ce cas présent. Voilà. Le président a dit ça oui ou alors ben nous on n'a pas trouvé que tout c'était forcément très bien placé dans les choix qui avait été fait, mais enfin bon c'est une vision particulière des, enfin là en tout cas, les choses se passent moins bien paraît-il. Semble-t-il. alors cet amendement fait il touche aux compétences du préfet de police mais mais pas seulement en Île-de-France, en fait puisque vous le savez, il y a de nombreuses autres villes de France qui accueille les Jeux olympiques et que les mairies qui sont intégrés dans des communautés de Covid métropole ou autres épaissi dans dans plus forcément les pouvoirs de police de stationnement et de circulation. Aussi, afin de leur permettre de faire face aux conséquences de la flûte personne à la fois sur la circulation, mais aussi sur certains sites particulièrement vulnérables, il convient de semble-t-il de leur permettent de manière strictement limitée dans le temps de pouvoir limiter la circulation et le stationnement sur leur territoire je l'exemple de ma ville, Marseille. Il se trouve que Marseille accueille. Les épreuves de. Que les épreuves nautiques seront visibles gratuitement de la totalité du littoral. Marseillais qui est assez large et qui était déjà sur fréquenté au niveau automobile et au niveau touristique en période normale et que donc ça va et que cette zone là étaient également le parc national des Calanques et qui les liait de biodiversité fragile et donc la ville de Marseille aimerait bien pouvoir disposer de ce pouvoir pour réglementer la circulation et le stationnement uniquement pendant la période des Jeux olympiques. vous voulez pendant le temps limité aux Jeux olympiques, que les maires puissent reprendre la compétence de stationnement du pouvoir de police de stationnement qui a été transférée aux EPCI. C'est une procédure qui est complexe, et ensuite votre amendement ne cerne pas vraiment quelles sont les communes qui sont concernées. Donc il manque d'opérationnel militer, c'est pour ça que nous émettrons un avis défavorable. Merci madame la ministre. Ma vie. Monsieur le président. Défavorable. Donc un double avis défavorable sur. Cet amendement. Je vais le soumettre aux voix qui est pour. Qui est contre. Qui s'abstient. Il n'est pas adopté. Amendement l'article 19. Madame la rapporteure. Monsieur le président, là au Sénat nous n'aimons pas beaucoup les ordonnances et en tout cas pas les non plus les les projets de loi d'habilitation. C'est pour ça que je vous propose. Une réécriture de l'article 19 qui concerne l'extension des dispositions du projet de loi à l'Outre- mer de manière à ce que ces dispositions soient inscrits en dur en dur dans le texte. Madame la Ministre. Elle dit fait avis favorable Monsieur président. Un avis favorable. Donc nous allons voter sur cet amendement qui vaudra. Vote sur l'article puisque enfin s'il est adopté. Parce que c'est une réécriture globale de l'article. Donc il est pour. L'amendement présenté par Madame la rapporteure avec un avis favorable du gouvernement. C'est contre. Qui s'abstient il est adopté. Donc l'article 19. Adopter ainsi rédigé. Et le dernier amendement un amendement sur l'intitulé du projet de loi monsieur Oui, merci Monsieur le Président. C'est un amendement sur l'intitulé puisqu'en fait. Nous pensons que une bonne partie de ce texte n'a pas grand chose à voir avec les Jeux olympiques pendant tous nos débats nous avons. Augmenter la répression compte Les Échos activistes. Nous avons augmenté la répression compte les supporters et surtout nous ne sommes lancés dans une nouvelle expérimentation de la vidéosurveillance. Automatisée donc de au nom des JO. Nous avons légiféré enfin surtout vous avez légiférer pour faire reculer nos droits et libertés. Vous avez décidé d'aller toujours plus vite pour jouer aux apprentis sorciers avec nos libertés publiques vous avez décidé d'aller toujours plus haut dans le recul des droits au nom du marché global de la sécurité, vous avez décidé les plus fort dans la société de surveillance en faisant des Françaises et des Français les cobayes d'une expérience sécuritaire siècle, ah les JO à Paris, c'est une fois par siècle nous a dit le ministre de l'Intérieur, il fallait comprendre ici comme une opportunité pour lui d'd'aggraver la situation. Il en a donc profité pour nous faire basculer dans le siècle de la surveillance globale privée et automatisé. Je vous propose donc de rester cohérent avec nos débats en renommant ce projet de loi en cohérence avec ce qui a été voté ici et en actualisant la devise olympique plus vite, plus haut, plus fort dans la surveillance, le contrôle et la répression. Je vous remercie. Madame la rapporteure. Merci monsieur le président, ce sera un avis défavorable sur cet amendement Mandement pardon, plein d'esprit mais qui porte un jugement de valeur que je ne partage pas sur le projet de loi. Nous préférons rester. Au titre que nous avons modifié en commission. Madame la Ministre. Même avis même avis. On a essayé de se centrer sur l'essentiel d'apporter les. Les garanties, la protection des droits et libertés et d'arriver à un texte qui est utile et équilibrée, mais je voulais. Néanmoins remercier sincèrement le le sénateur dessus pour son investissement sur ce texte et nos échanges qui l'avait précédé. Monsieur broyés. Je veux profiter de cet amendement taquin de de mon collègue Thomas Dossus. Pour rappeler que les. Le groupe écologiste a défendu avec vigueur l'intérêt de ces Jeux olympiques, au sens où ils représentent un espace de fraternité, une rencontre de la jeunesse du monde mais a souhaité aussi en préserver finalement l'esprit qui était celui de ses initiateurs et ça me permet de faire une page de publicité pour ma belle communes d'Arcueil en rappelant à tous ceux qui sont ici que c'est le sept mars 1880 ce que le père Didon prieur du collège Albert Legrand à Arcueil a donné la devise situs Altice fortune. À cet établissement de Dominicains situé sur le territoire d'Arcueil, grand ami de Coubertin. Il portait avec lui une vision éducative du sport.

Il était moderne de considérer que le sport, l'éducation physique était une constituante de l'activité éducative dans son ensemble. Voilà alors c'est un peu par mémoire au père Didon par mémoire à la caravane qu'il organisa pour les premiers Jeux olympiques des collégiens d'Arcueil en direction d'Athènes que je soutiendrai l'amendement de mon collègue dessus même si attaque hein pour dire qu'au fond ce qui comptera malgré tout dans ces Jeux olympiques, c'est le rassemblement de cette jeunesse la fonction éducative du sport, le sport a des vertus mais des vertus qui s'enseigne et souhaitons qu'il ne serve pas à d'autres usages que les meilleurs usages qui nous permettent de faire. Monsieur Breuiller pour ce rappel historique ouais lié à votre Cherville d'Arcueil. Nous allons voter sur l'amendement. 70. Avec un double avis défavorable qui est pour. Qui est contre. Qui s'abstient. N'est pas adopté. Donc nous avons terminé l'examen. Des armes. De ce texte. Je vous rappelle que les explications de vote et le vote par scrutin public sur l'ensemble du projet de loi se dérouleront lors de notre prochaine séance le mardi 31 janvier à 14h 30. Mais, chers collègues par lettre en date de ce jour, le gouvernement sollicite du Sénat l'inscription à l'Ordre du jour du mardi 7 février après-midi des conclusions de la commission mixte paritaire sur le projet de loi relatif à l'accélération de la production d'énergies renouvelables. Nous pourrions inscrire l'examen de ces conclusions après le débat sur le thème automobile tout électrique 2035 est-ce réalisable. Le délai limite pour les inscriptions de parole serait fixée au lundi 6 février à 15h. Y a-t-il des observations. Je n'en vois pas. Il en est ainsi décidé. Monsieur le président. Je voulais juste. Vous demander le, l'autorisation de vous remercier, mesdames les rapporteurs. Monsieur le rapporteur. Mesdames et messieurs et vous dire c'était un peu un baptême du feu pour moi mais j'ai eu vraiment beaucoup de, de plaisir à cette intensité à ces échanges avec vous dans l'attente du vol solennelle Mardi prochain. Je crois qu'on a. Eu des bons échanges utiles qui ont pu améliorer là où c'était nécessaire ce ce projet et je voulais sincèrement vous remercier de. Ces deux après-midi et de la soirée d'hier soir. Merci infiniment. Merci, madame la Ministre. Je vais donc levé la séance et on se retrouvera mardi prochaine séance donc mardi 31 janvier à 14h 30 pour les explications de vote, des groupes Sur solennel sur le projet de loi relatif aux Jeux olympiques et paralympiques de 2024. La séance est levée.